Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons analysé le projet de budget pour 2020

Rappelons que ce budget nous est présenté au terme d'une année marquée par le volontarisme du Gouvernement en matière d'aide publique au développement. Ainsi, la France a accordé une place centrale à la politique de développement lors du G7 qu'elle a présidé en août dernier, ou encore lors du G20 qui s'est tenu au Japon en juin dernier. Ces deux rendez-vous internationaux ont permis de réaffirmer notre attachement aux objectifs de développement durable et à la place centrale de l'Afrique dans notre aide. En premier lieu, le projet de budget pour 2020 poursuit la montée en charge des moyens budgétaires en faveur de l'aide publique au développement, même si l'essentiel de la hausse interviendra après 2020. Les autorisations d'engagement de la mission s'élèvent à 7,3 milliards d'euros, soit une hausse très importante, de près de 63 %. Les crédits de paiement s'établissent à 3,3 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 7 % par rapport à 2019. La forte progression des autorisations d'engagement résulte en réalité du cycle de reconstitution des ressources de plusieurs fonds et organisations multilatéraux en 2020, en particulier l'Association internationale de développement (AID), le Fonds vert pour le climat (FVC) et le Fonds africain de développement

Le produit des taxes affectées au développement est stable, à hauteur de 738 millions d'euros. À cet égard, le projet de loi de finances pour 2020 est marqué par une évolution notable. La taxe de solidarité sur les billets d'avion et le surplus de recettes affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf). Cette mesure a fait l'objet de vifs débats en séance publique, mais je tiens à rappeler l'importance de la sécurisation des ressources du Fonds de solidarité pour le développement auquel le produit de cette taxe est affecté. Nous avons un motif d'inquiétude concernant le programme 852 du compte de concours financiers, qui recouvre les crédits liés aux restructurations de dettes accordées par la France.

Après plusieurs auditions, il a semblé aux rapporteurs spéciaux que ce budget était encourageant pour atteindre l'objectif fixé par le Gouvernement. En effet, comme nous l'avons indiqué en commission,

sur les dispositions envisagées en la matière, en particulier sur le comité de pilotage que vous avez instauré voilà quelques semaines ? Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les quelques réflexions que m'inspire ce projet

comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, accordent presque la totalité de leur aide publique au développement sous forme de dons. Cette spécificité française entraîne un décalage entre la liste des pays que nous définissons comme prioritaires

-en autorisations d'engagement pour concrétiser cette promesse. Toutefois, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une réduction des ressources permettant à l'AFD d'accorder des dons, à hauteur de 594 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 35 millions d'euros en crédits de paiement. À l'inverse, la capacité de l'Agence à octroyer des prêts progresse légèrement. Les auditions que nous avons effectuées ont mis en évidence la volonté de revaloriser le rôle des ambassades dans le versement de subventions. Dans cette perspective, les crédits des fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) ont progressé de 36 millions d'euros. Ce choix suscite des interrogations de notre part, car la masse salariale des réseaux consulaires et diplomatiques est appelée à se contracter dans le cadre de la réforme de l'État à l'étranger. Les ambassades auront-elles les moyens d'absorber cette charge de travail supplémentaire ? La déconcentration de cette enveloppe ne risque-t-elle pas d'entraîner un effet de saupoudrage ? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment les ambassadeurs mèneront à bien cette nouvelle mission tout en poursuivant un objectif de réduction de leur masse salariale ? Cette perspective pose question sur les relations futures entre l'AFD et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

la commission des finances propose le rejet des crédits de la mission « Aide publique au développement ». Indépendamment de la question de l'évaluation de cette politique publique, les échanges nourris qui ont eu lieu en commission traduisent un certain malaise concernant les principaux bénéficiaires de notre aide publique au développement, en particulier la Turquie. La commission des finances s'est exprimée clairement en faveur d'une plus grande transparence dans l'allocation des crédits et de la mise en oeuvre d'un pilotage clair de cette politique publique. La coexistence de deux ministères de tutelle, d'acteurs étatiques, non étatiques, de l'opérateur pivot qu'est l'Agence française de développement, participe certainement d'une certaine confusion. Je vous remercie,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères partage nombre des préoccupations qui viennent d'être exprimées. Clarification de la stratégie et du pilotage, renforcement de l'évaluation, priorité à l'Afrique : tels sont nos principaux sujets d'intérêt pour l'année à venir, comme vous le savez, monsieur le ministre. matière de pilotage et de stratégie, nous notons avec satisfaction la volonté du ministère de réinvestir cet enjeu politique majeur. Nous pouvons nous féliciter de disposer d'un opérateur puissant pour notre action extérieure, mais il est impératif que sa stratégie reste alignée sur celle qui est définie par le Gouvernement et le Parlement.

il est essentiel que nous mettions en place un dispositif permettant au Parlement de co-définir le programme d'évaluation de la nouvelle instance et de demander au Gouvernement de s'exprimer devant nous sur les résultats obtenus. Je vous remercie, monsieur le ministre, de nous dire où en est votre réflexion

Or les besoins restent immenses, notamment dans le domaine de l'énergie, comme nous avons pu le constater la semaine dernière lors d'un déplacement à Madagascar. Et je ne parlerai pas des pays du Sahel, où le taux d'électrification n'atteint même pas 30 %. en matière d'aide au développement, qui se concrétise par l'augmentation des crédits alloués au Partenariat mondial pour l'éducation, est certes une bonne nouvelle. Il est en effet essentiel d'offrir un meilleur avenir aux enfants et aux jeunes d'Afrique subsaharienne,

Enfin, vous me permettrez de vous interroger sur un aspect technique de la coopération décentralisée, dont vous connaissez l'importance, notamment dans les territoires sensibles. Cette aide se trouve contrainte dans la limite du 1,2 % d'augmentation des budgets de fonctionnement, alors qu'il s'agit souvent de financements extérieurs. Je vous remercie, sur cette question également, des précisions que vous pourrez nous apporter.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'aborderai tout d'abord la situation d'Expertise France, tant la présence dans le monde de l'expertise française est un outil essentiel d'influence, notamment en Afrique, où nous risquons de passer au second plan par rapport à nos partenaires allemand et britannique.

En effet, l'intégration au groupe AFD est tout sauf une solution miracle : il faut notamment éviter que ne s'installe une relation exclusive avec l'Agence, qui priverait Expertise France de son accès à l'expertise des différents ministères et la ferait dépendre d'un

Il est question, semble-t-il, d'un rattachement de la future commission indépendante d'évaluation à la Cour des comptes. Nous nous interrogeons sur cette perspective. Le modèle britannique, que nous avons étudié lors d'un déplacement à Londres, nous paraît nettement plus pertinent

mais à condition qu'il y ait synergie, et non contradiction, avec notre action bilatérale. À cet égard, monsieur le ministre, sommes-nous au Sahel sur la même longueur d'onde que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ? De même, on sait que le Fonds mondial, auquel nous venons encore d'augmenter notre contribution, n'agit pas suffisamment pour renforcer les systèmes de santé des pays africains. Allons-nous réussir à infléchir cette tendance ou ne ferons-nous que la pallier par notre aide bilatérale ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission « Aide publique au développement » connaît une hausse très substantielle de ses crédits, qui représenteront l'année prochaine 0,43 % de notre revenu national brut. Nous saluons cette progression, bien que nous regrettions l'écart qui se creuse avec la trajectoire nécessaire pour atteindre l'objectif présidentiel de 0,55 % du RNB en 2022- sans parler des 0,7 % fixés dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies. Au-delà de cette hausse générale, nous constatons que l'aide publique au développement (APD) de la France est marquée par un fort déséquilibre entre les prêts et les dons, au détriment des seconds. Cela nous distingue de nos voisins, qui insistent plus que nous sur la dimension dons de leur APD. Cette situation n'est pas sans conséquence sur notre action. En effet, elle entraîne un écart sensible entre les priorités que nous affichons, notamment géographiques- je pense évidemment à l'Afrique -, et la réalité de notre action.

Dans l'attente d'éclaircissements à ce sujet, nous réaffirmons notre souhait que la hausse prévue des moyens accordés à l'APD inclue un rééquilibrage en faveur des dons. Par ailleurs, nous constatons que l'augmentation des crédits de la mission est particulièrement marquée en ce qui concerne la coopération multilatérale, principalement en autorisations d'engagement. Cette tendance résulte notamment de la hausse de la contribution de la France à plusieurs fonds multilatéraux, tels le Fonds vert pour le climat et l'Association internationale de développement. Il est important que la France participe à ces mécanismes internationaux en faveur des pays moins avancés, et nous y souscrivons. Cependant, nous constatons que ces autorisations d'engagement supplémentaires contrastent avec le recul de celles qui

En réduire l'ampleur est donc particulièrement regrettable, car nous pensons que l'APD française doit être pleinement intégrée à la politique étrangère de notre pays. De ce point de vue, la conditionnalité de l'aide, dans un cadre réglementaire strict, ne devrait pas être un tabou.

Plusieurs pays, plusieurs régions du monde sont en proie à des déséquilibres qui laissent craindre l'émergence, dans un futur proche, de situations contraires à nos intérêts. Il est donc essentiel d'agir de manière efficace, dès maintenant.

dans sa constitution, car associant positivement les commissions des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. Face à la dure réalité du terrain, nous avons pu nous rendre compte de l'action de la France à partir des projets présentés et menés par l'AFD

des affaires étrangères, Jean-Pierre Vial et Marie-Françoise Perol-Dumont : il est grand temps que soit précisé l'agenda du projet de loi d'orientation et de programmation relatif à l'aide publique au développement. La nature et l'efficacité de notre action dépendent des deux grands équilibres qui structurent le fonctionnement de l'APD : l'équilibre entre les dons et les prêts et l'équilibre entre l'aide multilatérale et l'aide bilatérale. Nous espérons que le futur texte, si nous en sommes saisis un jour,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2020 marque une nouvelle étape dans la remontée en puissance de notre politique d'aide au développement.

Les ressources extrabudgétaires, issues de la taxe sur les transactions financières et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, sont,

Je me réjouis également que le Fonds de solidarité pour le développement ait été recentré sur sa mission initiale : le financement de quelques fonds multilatéraux, dont le Fonds vert pour le climat. Sur le plan qualitatif, le projet de loi de finances est en phase avec les orientations du dernier Cicid. Plusieurs mesures budgétaires confirment le rééquilibrage de notre aide au profit de l'aide bilatérale sous forme de dons.

Un autre signe encourageant est l'augmentation importante des crédits destinés à la conduite de projets par les ambassades le fonds de solidarité pour les projets innovants. Cette excellente initiative soutient des projets de petite de petite ampleur, mais mis en oeuvre très rapidement et, j'espère, de façon efficace, à côté de la grosse machinerie que nous connaissons. Il convient de saluer aussi l'effort budgétaire en faveur de l'aide humanitaire et de la coopération décentralisée. Ces deux outils contribuent au renforcement du canal bilatéral de dons de notre aide. Il en va de même pour les contrats de désendettement et de développement, auxquels le projet de loi de finances consacre 42 millions En ce qui concerne l'aide multilatérale, il faut souligner le doublement de la contribution française au Fonds vert pour le climat qui prendra essentiellement la forme de dons. Voilà qui

Des inquiétudes se sont exprimées sur la baisse des autorisations d'engagement allouées aux dons-projets mis en oeuvre par l'AFD. Personnellement, je ne les partage pas. Je pense que le projet de loi de finances ne remet aucunement en cause les priorités thématiques et géographiques. L'effort budgétaire demeure très important. La discussion du très attendu projet de loi d'orientation et de programmation,

La commission indépendante d'évaluation qui devrait être mise en place sera chargée, notamment, de mesurer l'effet de l'APD sur les flux migratoires, le Gouvernement ayant récemment exprimé sa volonté de faire de cette aide « un levier au service de la politique migratoire ». affaires étrangères, le directeur général de l'AFD a déclaré, certainement à juste titre, qu'« une partie très significative de la réponse à la crise migratoire se trouve dans les pays d'origine, dans les pays de première destination et dans les pays de transit des migrants

lors de nos débats l'an dernier, nous avions tous conclu que nous attendions beaucoup d'une loi de programmation spécifique relative à l'aide publique au développement. Malheureusement, cette loi n'existe toujours pas

rassurer. Le seul objectif, martelé par le Président de la République, est d'atteindre, d'ici à la fin du quinquennat, 0,55 % du PIB consacré à l'aide publique au développement.

Bien évidemment, certains jeux d'écriture pourraient permettre de gonfler artificiellement le budget. Je pense tout particulièrement au recours accru aux fonds inscrits, mais bloqués. Cela suffira-t-il ? Je ne le pense pas. Il est urgent de redéfinir cette mission budgétaire. Tout d'abord, en augmentant massivement les crédits inscrits, sans se contenter de promesses. Ensuite, en réformant la taxation affectée à l'aide publique au développement.

Monsieur le ministre, nous avons dans ce domaine un certain désaccord : je ne conçois pas l'APD comme un outil conditionné aux bénéfices à en attendre pour notre pays.

le ruissellement, si cher à notre gouvernement, creuse toujours les inégalités chez nous : comment ne produirait-il pas les mêmes effets dans les pays en développement ? Compte tenu de ces observations, monsieur le ministre, nous voterons contre les crédits

mais elle recouvre bien d'autres aspects. En particulier, elle est l'un des outils majeurs de notre politique internationale : à travers elle, nous favorisons la diffusion de nos valeurs et nous servons nos intérêts. Une action menée dans un pays a des répercussions dans les autres, y compris en France. Ceux qui ne le comprennent pas voient cette aide, au mieux, comme une variable d'ajustement et, au pire, comme de l'argent jeté par les fenêtres. cette aide est un investissement, dont les retombées dépassent la seule sphère économique. De fait, elle est aussi une aide publique à la construction de la paix. Le travail est immense ... On s'en rend compte en regardant les missions de l'AFD au Sahel et dans les autres zones prioritaires.

brut. Nous nous rapprochons ainsi de l'objectif de 0,55 % fixé par le Président de la République. Cette augmentation et la logique qui la soutient nous paraissent être des signaux positifs. nous regrettons que l'objectif de 0,7 % du RNB ait été abandonné. En effet, cet objectif résulte de nos engagements internationaux, issus des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies de 1970. le Gouvernement poursuit le réarmement de notre politique d'aide au développement, ce dont nous lui savons gré. Le bénéfice de cette aide n'est pas unilatéral : le pays qui dépense en retire aussi des avantages. C'est ce qu'a bien compris le Royaume-Uni, qui consacre 0,7 % de son RNB à l'aide au développement : personne ne croit qu'il s'agit d'une pure philanthropie ... Cet exemple illustre, d'abord, fait que le Royaume-Uni considère, malgré les difficultés qui pèsent sur lui, que ces dépenses lui sont utiles ; ensuite, que cet objectif peut être atteint. Le Royaume-Uni n'est pas seul à adopter une politique d'aide au développement forte. C'est aussi le cas de la Chine, très active en la matière, notamment sur le continent africain et en Europe de l'Est- les nouvelles routes de la soie se construisent à travers l'Eurasie. L'Inde nourrit une ambition similaire et souhaite faire émerger un projet, concurrent, de route de la liberté. L'aide au développement façonne l'avenir, politique ou économique. La France doit y participer activement, en ayant cet objectif à l'esprit. nous sommes très favorables à la logique que vous défendez : comme vous, nous pensons que la France doit être maîtresse des dépenses qu'elle engage. Le multilatéralisme, bien sûr, n'est pas à fuir ; mais le bilatéralisme est à privilégier, lorsque nous ne nous retrouvons pas dans les projets multilatéraux. Notre action doit servir les intérêts de la France ; elle doit être efficace. À cet égard, plusieurs points d'amélioration subsistent. nous pensons qu'il faut améliorer l'articulation entre les actions de l'État, des collectivités territoriales, des ONG et des entreprises ou fondations privées. Elles peuvent parfois se compléter utilement. S'agissant de la gouvernance, nous considérons que la prise de décisions en matière d'aide publique au développement ne doit pas être éclatée entre deux ministères et un opérateur : cette division conduit à multiplier les instances de coordination et amoindrit la lisibilité et l'efficacité de notre politique d'aide au développement. concerne les objectifs de l'aide au développement, nous nous réjouissons que la priorité ait été donnée à l'Afrique, car nous pensons aussi que c'est sur ce continent que les efforts de la France doivent porter. De grands défis sécuritaires sont à relever, mais nous savons aussi que de grandes opportunités s'y développent. L'Afrique de demain va surprendre le monde ! Nous souhaitons que la France participe à son essor et à son développement.

les ambassadeurs dans leur rôle de chefs d'orchestre de l'action française de développement sur le terrain. La volonté exprimée de mieux intégrer l'AFD au sein de l'« équipe France » du développement, au moment où ses engagements atteignent un niveau vertigineux, de plus de 12 milliards d'euros,

pas suffisamment pour renforcer les systèmes de santé ? Dans le même temps, les pays africains qui construisent leur système de santé voient leurs crédits diminuer

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais relayer les propos préparés par André Vallini. Le projet de loi de finances prévoit une hausse de 210 millions d'euros de la mission « Aide publique au développement » pour 2020. Cette augmentation est bienvenue, mais elle reste insuffisante si on la rapporte à la trajectoire nécessaire pour tenir l'engagement, pris par le Président de la République, de consacrer, d'ici à 2022, 0,55 % de la richesse de notre pays à l'aide publique au développement. En 2019, le Gouvernement a mis l'accent sur l'augmentation des autorisations d'engagement. Cette hausse doit non seulement se poursuivre en 2020, mais être accompagnée d'une hausse significative, elle aussi, des crédits de paiement pour permettre une mise en oeuvre effective des projets.

pas dans les mêmes proportions par rapport à l'APD globale, ce qui ne permet pas une accélération de la mise en oeuvre des projets. Actuellement, la crainte est que les 0,55 % du RNB- objectif fixé par le Président de la République -soient affectés à tout ce qui ne concerne pas directement l'aide

dans la mesure, notamment, où la part des prêts reste très importante, alors que ce sont les dons qui permettent de soutenir au mieux les pays les moins avancés, en particulier dans les domaines sociaux et éducatifs.

20 %, en décalage par rapport aux annonces du Président de la République. Ensuite, la politique migratoire de la France présente un risque de dévoiement de l'APD, qui doit avoir pour objectif la lutte contre la pauvreté, les inégalités et leurs conséquences. Vouloir en faire un levier pour une autre politique revient à l'instrumentaliser au profit d'enjeux qui ne devraient pas lui être associés. Par ailleurs, comment ne pas s'interroger sur la confirmation de financements à certains pays- ce point a été évoqué précédemment -tels le Brésil ou la Turquie ? Comment justifier ces choix, au moment où le Président de la République a affirmé, à bon droit, vouloir concentrer prioritairement notre aide sur l'Afrique ? Compte tenu de la progression rapide des moyens qui lui sont consacrés, se pose la question de l'évaluation de l'aide publique au développement. Or, dans le projet de loi de finances pour 2020, les crédits dédiés à l'évaluation restent modestes, et aucune enveloppe spécifique n'est prévue pour le fonctionnement de la nouvelle commission d'évaluation qui pourrait être créée par la future loi d'orientation que nous attendions en 2019, et qui devrait arriver en 2020. Il devient donc urgent, dans le cadre de ce futur texte, de préciser les choix du Gouvernement en matière d'évaluation. le Royaume-Uni a adopté une loi fixant l'aide publique au développement à 0,7 % de son RNB et a créé, parallèlement, un dispositif d'évaluation avec un organisme dédié qui permet de rendre des comptes à la commission parlementaire chargée du développement. Sur ce point, je rejoins mon collègue Richard Yung : nous souhaitons qu'il en aille de même dans la prochaine loi d'orientation et de programmation. Sous réserve des critiques que je viens de formuler, et pour encourager le Gouvernement à aller plus loin et plus vite encore, nous voterons les crédits

si l'extrême pauvreté a reculé au cours de ces trente dernières années, notamment sous la pression des huit objectifs du millénaire pour le développement, les bouleversements qui agitent aujourd'hui notre monde nous invitent à rester vigilants sur cette évolution. En effet, aux fractures anciennes, qui avaient conduit au déséquilibre économique entre le Nord et le Sud, s'en ajoutent de nouvelles liées au changement climatique qui entraîne des déplacements massifs de populations. La crise migratoire qui a frappé l'Union européenne à partir de 2015 nous le rappelle : ce qui se passe là-bas n'est pas sans conséquence ici. La question du développement nécessite donc une action collective forte. En tant que cinquième contributeur, À cet égard, je rappellerai que notre pays a accueilli des annonces très importantes en matière d'aide au développement lors du G 7 qui s'est tenu à Biarritz, annonces qui, je l'espère, seront de nature à amplifier la remobilisation des États après le creux résultant de la crise financière de 2007-2008. Je salue également l'ambition que le Président de la République a affichée au début de son mandat et qu'il a réaffirmée depuis, à savoir porter l'aide publique au développement à 0,55 % de notre revenu national brut d'ici à 2022, sous réserve que ce cap soit atteint. Je me réjouis que la mission que nous examinons s'inscrive dans cette trajectoire volontaire. Les rapporteurs accordent d'ailleurs une confiance, certes prudente, mais réelle, à l'atteinte de l'objectif de 0,47 % du RNB.

La mission comporte une augmentation de la capacité de l'Agence à accorder des prêts à l'étranger grâce à une hausse des crédits de bonification des prêts de l'ordre de 1,1 milliard d'euros en autorisations d'engagement pour 2020.

ce débat sur le rapport entre les dons et les prêts, nous connaissons la conséquence de la prédominance des prêts : elle bouscule la définition des priorités, en ce qu'elle tend à exclure les pays les plus pauvres et les plus fragiles. À l'inverse, les grands émergents, dont le niveau de développement est assez élevé et qui bénéficient de prêts faiblement concessionnels, se voient ainsi bien soutenus par l'aide publique au développement. C'est pourquoi, sans remettre en cause les projets dans des pays qui participent de l'influence française dans le monde, il est toutefois urgent de redéfinir nos priorités. Aussi, nous attendons avec impatience l'examen par le Parlement du prochain projet de loi d'orientation et de programmation- vous l'avez confirmé, monsieur le ministre, Dans cette perspective, je souhaite d'ores et déjà évoquer quelques pistes tirées des enseignements du dernier rapport de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Ce document, mes chers collègues, soulève le manque d'efficacité de l'aide extérieure des contributeurs, qui ne ciblerait pas suffisamment leurs priorités de développement. Est-il normal, en effet, que dix pays sur quarante-sept captent 70 % de l'aide mondiale, parmi lesquels l'Angola qui va passer au statut de pays en développement en 2021 ? en 2021 ? Pourtant, une évidence demeure : c'est en Afrique que sévit la plus grande pauvreté, ce qui nous invite à réaffirmer son caractère de zone géographique prioritaire, s'agissant en particulier des pays les moins avancés.

Sans sous-estimer la persistance de grands défis sanitaires, on peut aussi relever que le soutien est en grande partie concentré sur l'éducation et la santé, à hauteur de 45 % du total de l'aide mondiale, alors que les infrastructures économiques, qui créent les emplois, n'en captent que 14 %. Enfin, il serait également souhaitable de bien évaluer la façon dont est canalisée notre aide sur place, afin que ne soient pas financées des multinationales avec de l'argent public. Je prendrai un exemple : les dons qui bénéficient à des cimentiers nationaux de pays d'Afrique francophone, cimentiers qui sont en réalité reliés au sein d'une multinationale, conduisent ces groupes à abaisser leur coût du travail au détriment d'entreprises vraiment locales. Toutes ces observations me conduisent à répéter que la remontée en puissance de l'aide publique au développement est indispensable, à condition de redéfinir clairement les orientations de celle-ci. Mes chers collègues, cette mission ne recouvre pas tout l'effort financier que nous consacrons au développement, mais elle est le reflet d'une dynamique entamée depuis quelques années, et dont on peut se réjouir. Le RDSE soutiendra bien entendu ce budget qui reflète une politique à laquelle adhèrent 79 % de nos concitoyens, bien conscients des enjeux qu'elle recouvre. En effet, et pour reprendre les mots de l'ancien président François Mitterrand, exprimés devant les Nations unies le 1 septembre 1981 : « La solidarité pour le développement [ ...] m'apparaît tout à la fois comme la clé de notre avenir commun et une nécessité pour chacun. » La parole est à M.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen du projet de loi de finances est un moment de vérité comptable et politique. La question qui nous est posée est la suivante : les crédits pour 2020 sont-ils à la hauteur des ambitions de la France sur la scène internationale ?

Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur la nature de l'aide publique au développement. Force est de constater que la part de l'aide directe a reculé au profit de l'aide sous forme de prêts en vertu de choix stratégiques étonnants.

alors qu'on impose des normes de traçabilité à tout va sur le territoire national, il est déroutant de constater qu'une banque publique française peut aider à coups de centaines de millions d'euros l'investissement dans un pays où l'échelle des valeurs est inversée. d'aides, alors même que la politique de M. Erdogan a pour incidence la résurgence de l'État islamique contre lequel nous sommes engagés au Levant et en Afrique. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, c'est au fléchage de l'aide que nous réagissons. Il est aux antipodes de la politique que vous menez, et pour laquelle vous oeuvrez sans relâche à la tête de votre ministère. J'en viens maintenant au point névralgique de l'APD française : son pilotage. Sur ce sujet, mon groupe soutient totalement la démarche du président Cambon et du rapporteur pour avis Jean-Pierre Vial qui appellent à une nouvelle relation avec l'administration, à sa responsabilisation et au retour à un véritable pilotage politique par le Gouvernement et le Parlement. C'est aussi de la tutelle des opérateurs de l'aide au développement qu'il s'agit. L'AFD dépend de Bercy. Néanmoins, pour tout ce qui concerne l'aide au développement, l'Agence et sa direction ne peuvent se substituer aux décideurs politiques.

Ce continent est menacé par l'islamisme extrémiste et a du mal à gérer sa croissance démographique exponentielle. Il représente un défi à l'échelle de la planète. J'aborderai maintenant l'importance de l'évaluation. Aucune politique ne peut se soustraire au contrôle. Sans évaluation, comment savoir si une politique doit être reconduite ou non ? Au moment où la réduction des dépenses publiques et les réformes touchent au coeur les Français, nous devons en permanence être animés par le souci de l'efficacité de chaque euro investi. investi. Avant de conclure, je souhaite revenir sur ce qui est devenu une très mauvaise habitude de Bercy, à savoir le détournement des produits des taxes, pourtant conçues pour alimenter des crédits de missions. C'est le cas de la taxe de solidarité,

mais au nom d'une volonté affichée de transparence et d'un meilleur pilotage politique. Nous souhaitons un retour à une politique cohérente avec notre diplomatie. Je sais que les travaux que vous engagez avec notre commission des affaires étrangères iront dans ce sens, mais nous voulons signaler la situation. La parole

de notre politique étrangère. Elle nous permet d'agir de façon concrète sur le terrain pour inscrire dans la durée nos efforts de gestion des crises, pour lutter contre les inégalités mondiales, pour protéger les biens communs que sont la planète, la culture et la santé des populations.

madame Perol-Dumont, qu'une partie de ces FSPI permet de financer des acteurs qui mobiliseront les financements ainsi déconcentrés. Toujours dans le cadre de notre aide bilatérale, l'aide humanitaire

nécessite. Quant aux moyens de l'AFD, ils vont de nouveau augmenter au titre de l'aide-projet avec 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement et une augmentation de 148 millions d'euros en crédits de paiement. que les normes de calcul de l'aide publique au développement se font en fonction des crédits de paiement, et non pas des autorisations d'engagement- c'est une précision tout à fait essentielle dans l'appréciation du projet budgétaire que je vous présente aujourd'hui. Je souhaite également que nous allons augmenter les fonds soutenant la société civile, avec un dépassement du seuil de 100 millions d'euros pour la subvention relative aux dons aux ONG mise en oeuvre par l'AFD, et que nous allons

s'agit de l'un des principaux opérateurs de notre politique de développement. Très bien ! En amont, c'est-à-dire en année n-1, mes services réalisent à ma demande un cadrage des secteurs prioritaires d'emploi du don-projet de l'AFD en pleine cohérence avec le Cicid.

nous ne signons pas un chèque en blanc en début d'année à l'AFD. C'est l'État qui fixera, sous mon autorité, les objectifs et les critères d'emploi des subventions et les orientations des prêts en pleine cohérence avec notre politique extérieure. En cours d'année, je tiendrai un conseil d'orientation stratégique de l'AFD avec l'ensemble des ministères concernés. Cette enceinte était en sommeil depuis 2011. Le prochain conseil se réunira dès le début de l'année J'ai par ailleurs souhaité que se tienne désormais un comité de pilotage plus restreint à mon niveau, avec le directeur général de l'AFD et l'un de mes collaborateurs tous les deux mois. L'objectif est simple réaliser des points d'étape réguliers sur l'activité de l'AFD et s'assurer que les résultats attendus sur le terrain sont au rendez-vous. Ce nouveau cycle a été inauguré il y a quelques jours. Ce pilotage politique de l'AFD ne doit pas seulement se faire à Paris. Il doit aussi se faire sur le terrain. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer considérablement le rôle de l'ambassadeur, qui doit être le pilote unique de l'équipe France, rassemblant l'ensemble des acteurs qui travaillent au sein de l'ambassade ou auprès des opérateurs. Très bien ! Concrètement, l'ambassadeur doit être en position d'assurer la pleine cohérence entre tous les instruments de notre politique, qu'ils soient à la main du poste ou d'opérateurs comme l'AFD. Nous allons mettre en place à cette fin un conseil local du développement présidé par l'ambassadeur qui lui permettra d'orienter tous les efforts- de l'État, de l'AFD et des ONG françaises -sur un même territoire. Très bien ! Les objectifs globaux seront précisés dans le projet de loi de programmation, et les initiatives que je prends seront aussi inscrites dans ce texte.

elle éloigne de la réelle APD les pays qui en ont le plus besoin. Les principaux bénéficiaires sont la Colombie, le Maroc, l'Indonésie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ces pays ont certes besoin d'être accompagnés dans leur développement, mais ils ont comme point commun une économie suffisamment développée pour leur permettre d'être solvables.

Le budget consacré à l'aide publique au développement a augmenté de plus de 3 milliards d'euros par rapport à la loi de finances pour 2019 ; on ne peut que s'en réjouir. Pour autant, il privilégie l'aide économique et financière- donc une logique de prêts et non de dons -, et les aides multilatérales, ainsi que les grands bailleurs internationaux au détriment d'une aide bilatérale classique fondée sur la solidarité et l'aide-projet. pour 2020 prévoit d'ailleurs une baisse de 520 millions d'euros des autorisations d'engagement du don-projet par rapport à 2019. amendement vise à flécher 100 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires vers l'action n° 02, Coopération bilatérale, au sein du programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », et à réduire de 100 millions d'euros les crédits de paiement de l'action n° 01, Aide économique et financière multilatérale, au sein du même programme. Il a donc pour objet d'augmenter les crédits de l'action Coopération bilatérale de 100 millions d'euros destinés à alimenter une aide publique au développement fondée sur la solidarité, et non sur la rentabilité des investissements.

Et quand je dis que je ne suis pas admiratif, je veux dire que nous sommes extraordinairement critiques : l'AFD dérape, l'AFD dérive ! On constate une absence totale de pilotage politique. Vous nous annoncez que

compliqués. L'AFD a toujours voulu voler de ses propres ailes, mais à chaque fois que le Gouvernement a été en mesure de faire respecter ses orientations politiques, cela n'a posé aucun problème.

Lepage. Cet amendement va dans le même sens. Le Président de la République a fixé des objectifs ambitieux pour l'aide publique au développement. Il a également souhaité que cette politique soit plus efficace et plus utile pour celles et ceux à qui elle est destinée. Le renforcement de la coopération au service du développement économique et du progrès humain exige une très forte mobilisation de la communauté internationale, qui associe, au-delà des États, tous les acteurs du développement, en particulier les ONG. Ces dernières sont devenues au fil des années de véritables acteurs au coeur des enjeux du développement, nécessaires à la mise en oeuvre de notre politique.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

notamment sur les actions entreprises pour améliorer la situation économique des États faisant appel à leurs concours, ainsi que sur la position de la France au sein de ces organisations et sur l'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces organisations. La commission des finances estime que la plupart de ces informations sont déjà partiellement accessibles dans les rapports d'activité annuels du FMI et de la Banque mondiale. En outre, plutôt qu'une nouvelle demande de rapport annuel, la commission des finances considère qu'il revient au Gouvernement de remettre au Parlement, chaque année et en temps utile, le rapport de synthèse de la politique de développement et de solidarité, tel que le prévoit déjà la loi d'orientation et de programmation de 2014. Enfin, un doute subsiste quant à l'appartenance de cet article au domaine des lois de finances, tel qu'il est défini par l'article 34 de la LOLF.

La faiblesse des moyens accordés au programme 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », qui représentait 46 % des crédits de la mission « Santé », est principalement due à des mesures de périmètre, accompagnées de coups de rabot sur les dépenses d'intervention. L'effort de maîtrise des dépenses sur la mission « Santé » repose d'ailleurs uniquement sur le programme 204, dont les crédits ont diminué de 69 % depuis 2013, tandis que le programme 183 a vu ses crédits progresser de 27 % sur la même période. Dans ces conditions, en raison d'importantes mesures de périmètre, représentant une baisse de 266,1 millions d'euros et sur lesquelles je vais revenir, les crédits de paiement demandés au titre de la mission « Santé » pour 2020 s'élèvent à 1 143,5 millions d'euros. À périmètre constant, ce montant correspond à une baisse de 1 % par rapport à 2019. S'agissant des mesures de périmètre, je m'interroge sur leur bien-fondé. Elles consistent en effet en des transferts de crédits destinés à des opérateurs du budget de l'État vers la sécurité sociale. mouvements ne m'apparaissent pas suffisamment justifiés et ne peuvent uniquement être motivés par une clarification de la répartition des compétences entre l'État et la sécurité sociale, sauf à conduire à la disparition de la mission « Santé Les missions assignées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et à l'Agence nationale de santé publique (ANSP) ne relèvent pas, de prime abord, d'une logique contributive que suppose, pourtant, leur rattachement au budget de la sécurité sociale. Au-delà des questions de périmètre, je m'interroge sur l'efficacité même du programme consacré, je vous le rappelle, à la prévention. Les indicateurs de performance visant la lutte contre le tabagisme, la vaccination contre la grippe ou le dépistage du cancer colorectal suscitent des interrogations sur l'efficacité de la dépense publique en matière de prévention, tant les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je m'inquiète, en outre, de l'écart entre les ambitions annoncées par le Gouvernement en matière de santé et leur trajectoire budgétaire. Concernant le programme 204, je relève un effort de sincérité budgétaire dans deux dossiers- la Dépakine et Wallis-et-Futuna -qui vient répondre directement aux remarques formulées par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi de règlement pour 2018. Venons-en désormais à ce programme 183, consacré quasi intégralement à l'aide médicale de l'État, la fameuse AME. Le maintien au niveau de 2019 des crédits consacrés à l'AME, soit 934,4 millions d'euros, n'apparaît pas soutenable au regard de la progression de la dépense constatée en 2018-

de 46 % en montant et de 25 % en nombre de bénéficiaires depuis 2012. Les crédits prévus pour 2020 traduisent, de fait, une nouvelle sous-budgétisation de l'AME pour soins urgents 30 millions d'euros entre l'exécution de 2018 et la prévision pour 2019 et 2020. Cela aboutira inévitablement à une progression de la dette à l'égard de la Caisse nationale d'assurance maladie, déjà établie à 35 millions d'euros. La part croissante des dépenses d'AME dans le budget de la mission « Santé » tend à réduire celui-ci à une enveloppe de financement de ce dispositif. Son dynamisme, conjugué à une sous-budgétisation récurrente, incite à l'adoption de mesures structurelles, visant les modalités d'accès aux soins et le panier de soins, afin de limiter sa progression, de répondre à l'impératif de sincérité budgétaire et de garantir la soutenabilité de la

la mission « Santé » se trouve désormais confrontée à une véritable crise existentielle. Le basculement vers l'assurance maladie du financement de la plupart des agences responsables de notre politique sanitaire pose la question de la pertinence d'un programme 204 qui ne comprend plus, comme opérateur à part entière, que l'Institut national du cancer Or ce dernier a lui-même vocation à voir ses moyens reportés à terme sur le budget de l'assurance maladie. Faut-il comprendre, madame la secrétaire d'État, que le programme 204 disparaîtra bientôt J'en viens aux crédits du programme 183, « Protection maladie ». Pour 2020, il est prévu de consacrer un peu plus de 919 millions d'euros au financement de l'AME, un montant en diminution de 15 millions d'euros par rapport à 2019. Cette baisse, résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, tire les conséquences des mesures de restriction des conditions d'accès à certains soins pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État. Sur le plan de la sincérité budgétaire, la dépense d'AME semble désormais mieux maîtrisée. Les projections du Gouvernement se fondent sur une hypothèse globale de stabilisation du nombre de bénéficiaires en 2019 et 2020. Compte tenu du renforcement de la lutte contre l'immigration illégale, l'hypothèse d'un reflux du nombre de bénéficiaires à moyen terme n'est d'ailleurs plus à exclure. La commission des affaires sociales a réaffirmé néanmoins son opposition à la réinstauration d'un droit de timbre. Déjà expérimentée par le passé, cette mesure est inefficace : faute d'accès aux soins de prévention, les personnes en situation irrégulière se présentent effectivement aux urgences, avec une prise en charge dont le coût sera aggravé par leur état de santé dégradé. Le résultat, c'est un transfert de la charge sur le budget des hôpitaux. De même, notre commission s'inquiète des tentations de réduction du panier de soins de l'AME. Sur l'initiative du Gouvernement, les députés ont institué un délai d'ancienneté dans le dispositif de l'AME pour bénéficier de certains soins. Il serait utile, madame la secrétaire d'État, que vous nous précisiez le fonctionnement des mécanismes d'entente préalable entre l'assurance maladie et l'équipe médicale qui garantiront, je l'espère, l'accès aux soins lorsque l'examen clinique le justifie, même si la condition d'ancienneté n'est pas remplie. N'oublions pas, en effet, que seuls les soignants sont en capacité de définir le parcours de soins le plus pertinent compte tenu de l'état de santé du patient. Sous réserve de ces observations, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Santé ». Mes chers collègues, je vous rappelle

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous aurions pu adopter sereinement un budget stabilisé et sincère si le Gouvernement n'avait délibérément lancé et alimenté une séquence détestable sur l'aide médicale de l'État. Au lieu de cela, l'examen de la mission « Santé », cette année, est entaché par une polémique qui n'honore pas le parti présidentiel, à rebours des engagements pris par le Président de la République et du soutien apporté jusque-là par la ministre de la santé,

Ce mauvais feuilleton a démarré avec la dénonciation de la fraude, à grand renfort de fausses informations, la plus scandaleuse ayant été celle de femmes étrangères qui viendraient en France pour se faire poser des prothèses mammaires aux frais de l'aide médicale de l'État. Il a donc fallu attendre le rapport des corps d'inspection pour démentir, point par point, ces allégations. Non, le panier de soins de l'AME ne comporte pas de soins dit « de confort Il est plus réduit que celui des assurés sociaux et exclut les médicaments à faible service médical rendu, les médicaments princeps pour lesquels un générique existe, la PMA ou encore les cures thermales. Il ne comporte d'ailleurs pas de programme de prévention, comme des dépistages bucco-dentaires pour les enfants, alors même que davantage de soins préventifs reviendraient à mieux contenir les dépenses. Non, hormis quelques filières organisées contre lesquelles il faut bien entendu lutter, la fraude à l'aide médicale de l'État n'est pas massive. Elle est même marginale, trois fois inférieure, en ordre de grandeur, à la fraude à l'assurance maladie. Non, le problème de l'aide médicale de l'État n'est pas d'ordre financier.

Cette séquence fut donc lamentable et, malgré les démentis, le mal est fait. Ces polémiques alimentent préjugés et divisions. Que le Gouvernement le veuille ou non, il a nourri une nouvelle fois la remise en cause de l'ensemble du dispositif.

-dissimule au fisc 57 % de son chiffre d'affaires réalisé en France, on se dit que l'égalité devant la répression des fraudes n'est pas au rendez-vous.

le périmètre de ce programme est de nouveau notablement réduit avec le transfert des financements de deux agences clés : l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette trajectoire confirme les interrogations et inquiétudes que nous avions Quel avenir pour un programme 204 en pleine « crise existentielle », dans un contexte d'affaiblissement du pilotage et des outils de notre politique de santé publique par le ministère, au profit d'une concentration croissante au profit de l'assurance maladie ? Concernant des sujets aussi majeurs que le médicament, d'une part, et l'expertise et la prévention en santé publique, d'autre part, ces transferts doivent s'inscrire dans une stratégie claire et partagée avec la représentation nationale. Cela s'avère d'autant plus impératif que le lien de confiance s'est distendu entre nos concitoyens et la politique sanitaire. Oui, je rappelle que le chef de l'État n'avait pas cru utile d'inscrire la santé dans les thèmes du grand débat, mais les Français l'ont placée en tête de leurs préoccupations,

Affaiblissement du pilotage politique du ministère ou « étatisation » de l'assurance maladie ... Difficile, en tout cas, de saisir les tenants et aboutissants de cette orientation, s'agissant de politiques publiques qui appellent pourtant à une détermination sans précédent. Je m'en tiendrai à trois exemples. concerne la santé environnementale, dont les crédits sont rehaussés à hauteur de 40 % cette année. C'est très bien ! Rappelons toutefois que l'effet de cette hausse, en prévision du plan « Mon environnement, ma santé » annoncé pour avril prochain, est limité par la baisse de 20 % à laquelle il avait été procédé l'an passé.

La puissance publique, en matière de volontarisme politique et de financements, n'est malheureusement pas à la hauteur des enjeux. À cet égard, comment expliquer qu'en 2019 un président de la République puisse céder aux et décider, de lui-même, d'annuler une campagne de santé publique

financée à hauteur de 4,85 millions d'euros pour 2020. Les résultats encourageants publiés récemment par Santé publique France en matière de baisse des nouvelles contaminations appellent à redoubler d'efforts sur la prévention et le dépistage. Nous y reviendrons au Parlement. Madame la secrétaire d'État, la mission « Santé » ne résume ni ne porte à elle seule notre politique de santé. Heureusement ! Mais le Parlement ne devrait pas seulement être amené à constater quelques évolutions ; il devrait être pleinement associé au nécessaire travail de redéfinition du périmètre et du rôle du programme 204. Je ne peux que vous inviter à le faire. Très bien

cette mission « Santé » du projet de loi de finances a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières semaines, prise au coeur d'un débat sur l'immigration et l'accueil des demandeurs d'asile. Cette mission contient effectivement deux programmes. Celui qui est consacré à l'aide médicale de l'État reste au coeur des préoccupations, puisqu'il représente désormais 82 % des crédits de la Néanmoins, attachée aux questions de prévention, je commenterai d'abord les ressources allouées au programme 204. Ce programme est remanié dans son périmètre, passant de 7 opérateurs en 2015 à 2 opérateurs en 2020. Cette année, ce sont les dotations de l'ANSM et de Santé publique France qui sont transférées à l'assurance maladie.

Mais j'insisterai aussi sur deux autres sujets. D'une part, le taux de vaccination contre la grippe, qui tue encore 10 000 personnes chaque hiver, stagne chez les plus de 65 ans. Les mesures de simplification de l'accès à la vaccination décidées dans le plan « Ma santé 2022 » devraient, je l'espère, corriger cette

Il stagne, après une amélioration avant 2015. Encore plus de 12 % des prélèvements d'eau potable ne sont pas microbiologiquement conformes, et c'est sur les petits réseaux, de moins de 500 habitants, que cette non-conformité est significativement plus élevée. Cela peut nous interroger.

(CPP), qui jouent un rôle important dans l'accès précoce aux médicaments innovants. Nous saluons l'augmentation pérenne de leur budget à hauteur de 700 000 euros, qui permettra le financement de 14 équivalents temps plein supplémentaires. C'est une avancée, qui reste toutefois insuffisante pour permettre aux 39 CPP de fonctionner de manière continue. Mais nous ne manquerons pas de revenir plus en détail sur le sujet, lors de l'examen de la proposition de loi que je défendrai avec mes collègues Catherine Deroche et Yves Daudigny. J'en viens maintenant au programme 183, consacré presque exclusivement au financement de l'aide médicale de l'État, à hauteur de 934 millions d'euros, ce qui en fait, d'après le rapport conjoint de l'Inspection À titre personnel, ce n'est pas celui qui m'inspire le plus ! Face à de tels sujets, complexes et sensibles, j'aime à me rappeler les grands principes guidant ma réflexion : l'humanisme et le respect de la personne ; la protection de la santé publique ; la bonne gestion des deniers publics. un équilibre à trouver : ni trop, ni trop peu ... La commission des finances a déposé plusieurs amendements, afin de transformer l'AME en aide médicale d'urgence (AMU), de réduire le panier de soins et de créer un droit de timbre. L'AME est trop souvent considérée comme un élément de politique migratoire, alors qu'elle est un dispositif de santé publique. En accord avec la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, mon groupe, dans sa grande majorité, ne soutiendra pas ces amendements. S'agissant des modifications introduites à l'Assemblée nationale, nous prenons note des mesures visant à lutter contre la surconsommation et la fraude. Je partage la nécessité de combattre ces dernières, quand elles existent ! Les moyens de contrôle seront-ils toutefois suffisants ? Revenons-en à des termes budgétaires. Les dépenses au titre de l'AME, bien qu'en augmentation, ne représentent que 0,5 % des dépenses de l'assurance maladie. L'impact des dernières annonces sur le budget de la mission- soit 15 millions d'euros d'économies prévues -va dans le sens d'une maîtrise budgétaire, que nous saluons. Toutefois, veillons à ce que certaines de ces mesures, notamment l'allongement du délai d'accès, ne soient pas contre-productives, car des pathologies prises en charge avec retard nécessitent des traitements plus longs, plus lourds et plus coûteux. Une évaluation stricte et rapide de la mesure sera nécessaire. On peut effectivement regretter le peu de chiffres, de statistiques à même de nous éclairer dans notre réflexion, ce qui, souvent, est propre à ouvrir la voie aux fantasmes. Je terminerai en rappelant que les médecins continueront à exercer leur profession et à soigner les malades, tous les malades ! Faisons leur confiance pour apprécier, au cas par cas, les besoins de chaque patient ; il est indispensable de préserver cette marge d'appréciation des soignants, qui sont en première ligne. Voilà deux ans, à la même tribune, j'ai conclu en disant qu'il fallait se pencher sur le sujet avec pragmatisme et sans posture. C'est dans ce même état d'esprit, dans l'attente de quelques réponses sur le volet concernant la prévention et avec les quelques réserves émises que mon groupe, dans sa grande majorité, votera en faveur des crédits de la mission « Santé ». La

le montant global des crédits de la mission « Santé » ouverts pour 2020 s'élève à un peu plus de 1 milliard d'euros en crédits de paiement. Ce montant enregistre une baisse de 19 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2019,

Ce différentiel s'explique principalement par le transfert, de l'État à l'assurance maladie, du financement de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé et de l'Agence nationale de santé publique. Cette baisse s'explique également par les efforts financiers demandés aux opérateurs de santé dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. C'est un budget cohérent qui porte haut les engagements de la stratégie nationale de santé 2018-2022 et du plan Ma santé 2022. Il doit permettre de développer la politique de prévention, d'assurer la sécurité sanitaire et d'organiser une offre de soins de qualité pour nos concitoyens de l'Hexagone et des outre-mer. La mission « Santé » comprend deux programmes, que je détaillerai brièvement. Le programme 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », doit permettre d'améliorer l'état de santé général de la population. Son ambition est de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, mais également de prévenir et de maîtriser les risques sanitaires. Nous pouvons nous réjouir qu'un effort particulier soit apporté à la recherche sur le cancer : les chiffres de cette et les progrès encore limités. Un peu plus de 41 millions d'euros en crédits de paiement sont ainsi consacrés pour 2020 au financement de l'Institut national du cancer, chargé de la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Les crédits ouverts pour la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation connaissent, quant à eux, une forte augmentation. Ils s'élèvent pour 2020 à 25 millions d'euros contre un peu plus de 18 millions d'euros en 2019. Ces crédits permettront de renforcer le rôle et l'action de l'Institut national Les dépenses d'indemnisation des victimes de la Dépakine vont, par ailleurs, faire l'objet d'ajustements structurants afin d'accélérer le traitement, jusque-là complexe, des dossiers. Le dispositif d'indemnisation, dont la gestion est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a effectivement connu une montée en charge progressive au cours des dernières années. Les crédits seront ainsi portés à 53,6 millions d'euros pour l'année 2020. Le programme 183, « Protection maladie », agit en faveur de l'accès aux soins des publics les plus défavorisés et de l'indemnisation des victimes de l'amiante. Avec un budget global supérieur à 942 millions d'euros, il est inchangé par rapport à la loi de finances initiale pour 2019. Le programme 183 est consacré, pour l'essentiel, à l'aide médical de l'État, dont la gestion est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Permettez-moi, mes chers collègues, de m'attarder un instant sur ce dispositif. Autant le rappeler d'emblée, il n'est pas question, à mon avis, de supprimer l'aide médicale de l'État ! Heureusement ! Il n'est pas non plus question de supprimer le droit à l'assurance maladie pour les demandeurs d'asile, de revenir sur le panier de soins ou d'exiger une participation financière aux bénéficiaires à l'AME. Selon nous, rien dans ce budget ne vient remettre en cause les grands principes humanitaires, auxquels nous sommes tous attachés. Au cours des dernières années, le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de manière importante. Près de 300 000 personnes bénéficient du dispositif aujourd'hui. Cette hausse a entraîné un accroissement des dépenses de l'État en 2018, celles-ci s'élevaient à 848 millions d'euros, soit une hausse de 6 % par rapport à 2017. Ce constat a conduit le Gouvernement à s'interroger sur l'efficience du système, et sur ses éventuels abus. Un rapport de l'IGAS a proposé certaines améliorations. Nombre d'entre elles ont été intégrées au texte lors de son examen à l'Assemblée nationale, afin d'améliorer la gestion des demandes et de mieux réguler les dépenses de l'AME et des soins urgents. Ces améliorations concernent notamment la lutte contre les abus, qui se voit ici renforcée. Il est envisagé de conditionner la prise en charge de certaines prestations programmées et non urgentes, pour les bénéficiaires majeurs de l'AME, à un délai d'ancienneté. Les demandeurs devront désormais se présenter en personne à la caisse primaire d'assurance maladie pour déposer leur demande d'aide. Enfin, un délai de carence de trois mois est également évoqué pour les demandeurs d'asile souhaitant bénéficier de la protection universelle maladie. L'enjeu n'est pas ici de restreindre les droits des personnes migrantes, mais de réprimer les abus constatés dans le cadre de l'AME, et de permettre à ceux qui y sont éligibles d'en bénéficier pleinement. Lors de l'examen de ce texte en commission des finances, plusieurs amendements du rapporteur spécial ont été adoptés. Ils limitent, voire suppriment l'AME, en lui substituant une aide médicale d'urgence. Ce débat n'est pas nouveau. De telles propositions sont contraires à l'esprit de solidarité et d'humanisme qui anime notre groupe. Les raisons en sont nombreuses et elles ont été énoncées à de multiples reprises. La commission des affaires sociales, saisie pour avis, a d'ailleurs proposé d'adopter les crédits de la mission « Santé » sans modification. Pour ces différentes raisons, notre groupe votera les crédits tels qu'ils ont été proposés par le Gouvernement. Dans le cas contraire, il votera contre.

Comme cela a été dit par mes prédécesseurs, notamment par la rapporteure Corinne Imbert, que je tiens à remercier pour la qualité de son rapport, nous examinons les crédits d'une mission « Santé » très restreinte, ce que je déplore fortement. Le transfert de l'ANSM et de l'ANSP vers l'assurance maladie est non seulement un non-sens sur le fond, mais entraîne, pour la mission « Santé », et plus précisément pour le programme 204, une réduction à la portion congrue. La mission devient quasi fantomatique. Nous avons d'ailleurs déposé, pour la nouvelle lecture du PLFSS, demain, un amendement pour arrêter ce transfert.

Une nouvelle fois, comment ne pas être profondément choqué par l'attitude du laboratoire Sanofi, qui refuse de prendre ses responsabilités et d'indemniser les victimes de la Dépakine ? Pour notre part, nous sommes favorables à certaines pistes évoquées par la rapporteure. Comme souvent, madame la secrétaire d'État, vous allez répondre qu'une réflexion est en cours, mais, en tant que parlementaire, je suis preneuse d'informations, et je pense ne pas être la seule dans cet hémicycle. Le troisième point que je souhaiterais aborder porte sur les crédits liés à plusieurs actions, à savoir celle sur les traumatismes et les violences, celle sur la prévention des addictions, ainsi que celle en faveur de la santé mentale autant d'actions essentielles qui auraient besoin d'un soutien particulier de l'État. Je dois donc vous faire part de l'étonnement de notre groupe, quand il a constaté que ces actions ne bénéficient d'aucune augmentation de crédits par rapport à l'an dernier.

Comment ne pas regretter qu'il n'y ait pas de crédits supplémentaires pour créer de nouvelles unités de prise en charge globale du psycho-traumatisme ? Comment comprendre cette stagnation, après la formidable mobilisation du 23 novembre, qui a vu défiler plusieurs milliers de personnes dans toute la France, réclamant un milliard d'euros ? décalage entre les annonces du Premier ministre et la réalité budgétaire ! Personne, aucune association d'aide aux victimes, d'accompagnement des femmes victimes de violences, n'est dupe. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen de la mission « Solidarité, Dans le domaine des addictions, là aussi, nous nous étonnons que, malgré le lancement du plan gouvernemental en fin d'année 2018, nous retrouvions cette année exactement les mêmes montants. Enfin, nous faisons la même critique quant aux crédits consacrés à la santé mentale, car, là encore, pas un euro de plus n'est consacré à cette action, malgré la situation dramatique vécue par les établissements psychiatriques et les structures extrahospitalières. Enfin, j'en viens à mon quatrième point, l'AME.

Pourquoi alimenter de nombreux fantasmes autour de l'AME, quand seuls 38 cas de fraude ont été constatés l'année dernière, pour un préjudice d'à peine 500 000 euros, soit 0,06 % du montant total de l'AME ? Bien sûr, la loi doit punir les fraudeurs, mais avouez que c'est infinitésimal. Pourquoi ne pas montrer la même diligence à l'égard de la fraude patronale, qui s'élève à plusieurs milliards ? Madame la secrétaire d'État, au-delà de la baisse de crédits, c'est bien le fond de votre réforme qui est profondément choquant, puisque vous prévoyez non seulement de restreindre les conditions d'accès à l'AME, en créant un délai de carence pour accéder à la protection universelle maladie (PUMa), mais également de réduire la durée de l'AME de moitié pour les déboutés d'asile et les personnes sans-papiers. Tous les médecins que nous avons auditionnés s'opposent à ce genre de mesures restrictives, qui risquent de favoriser des épidémies et sont contraires au serment d'Hippocrate. Madame la secrétaire d'État, avec votre réforme, vous remettez purement et simplement en cause l'accès universel aux soins, en stigmatisant les personnes étrangères. vous rappelle que l'AME ne représente que 0,4 % des quelque 204 milliards d'euros de dépenses de soins. C'est un dispositif de santé publique, de prévention des maladies et des infections qui profite à toute la société, et ne relève en aucun cas du tourisme médical. Par son attitude, le Gouvernement, qui chasse sur les terres de la droite extrême, encourage une remise en cause toujours plus profonde de l'AME, notamment au moment de l'examen du PLF. Je souhaite m'adresser à notre collègue M. Joyandet et à une partie de la commission des finances ; je leur demande de renoncer à la suppression de près d'un tiers des crédits liés à l'AME, au droit de timbre et à la limitation du panier de soins, pour les raisons que je viens d'évoquer. Si ces amendements étaient maintenus, nous ne pourrions les voter, comme, je pense, bon nombre de mes collègues de la commission des affaires sociales, toutes sensibilités politiques confondues. Pour conclure, nous ne voterons pas les crédits de cette mission. La parole est à Mme Colette Mélot. Monsieur le président,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons à présent les crédits de la mission « Santé » du projet de loi de finances pour 2020, consacrée aux dépenses de santé non couvertes par le budget de la sécurité sociale. Cette mission regroupe deux programmes. Le programme 183 concentre 82 % des crédits ; il est essentiellement consacré au financement de l'aide médicale de l'État pour un montant stable de 934,4 millions d'euros, et au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le programme 204 rassemble un peu moins de 18 % des crédits de la mission ; il finance les actions de prévention, de sécurité sanitaire et d'amélioration de l'offre et de la qualité des soins pris en charge par l'État. L'enveloppe globale pour 2020 s'élève à 1,144 milliard d'euros en crédits de paiement, contre 1,422 milliard en 2019, soit une diminution de presque 20 %, très inégalement répartie entre les deux programmes. En effet, l'effort de maîtrise budgétaire repose essentiellement sur la révision du périmètre du programme 204, désormais réduit à peau de chagrin, après le transfert vers l'assurance maladie des crédits de financement de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé et de l'Agence nationale de santé publique. Les actions de ce programme ont connu une baisse de 69 % de leurs crédits depuis 2013, tandis que les dépenses finançant l'AME connaissent une hausse de 27 % sur la même période. Nous partageons les interrogations émises par le rapporteur spécial de la commission des finances, M. Joyandet, sur la place de ce programme au sein du budget de l'État et sur l'efficacité de la dépense au regard de ses objectifs de performance. En définitive, quelle est la priorité du Gouvernement en matière de prévention ? Les indicateurs proposés ont-ils démontré leur pertinence et l'efficacité des dépenses de prévention ? Le seul opérateur restant intégralement financé par cette mission est l'Institut national du cancer (INCa), dont les missions ont été élargies par l'adoption de la loi du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques. Aussi, la mission « Santé » du PLF pour 2020 tend à se résumer au financement de l'AME, sans doute le milliard le plus polémique de la dépense publique. Cette somme ne représente que 0,6 % de la dépense publique de santé en France, mais notre pays est l'un des plus généreux en termes d'accès au soin pour les étrangers en situation irrégulière.

Nous partageons l'avis du rapporteur spécial, qui dénonce une sous-budgétisation des crédits de l'AME consacrés aux soins urgents. Afin de maîtriser la hausse tendancielle des prestations, le Gouvernement propose notamment d'instaurer un délai d'ancienneté, de réguler l'accès aux soins non urgents et de renforcer les contrôles au stade de l'instruction des demandes. Il s'agit de vérifier la durée minimale de présence sur le territoire ouvrant droit à l'AME, fixée à trois mois, et d'effectuer des contrôles ciblés sur les soins les plus onéreux. La commission des finances souhaite aller plus loin. Elle propose d'instaurer un droit de timbre de 30 euros, de remplacer le dispositif par une aide médicale d'urgence de restreindre le panier de soins, afin d'harmoniser la couverture de soins offerte aux étrangers en situation irrégulière présents en France avec celle de nos partenaires européens, tels que l'Espagne, le Danemark ou encore l'Allemagne. Si nous soutenons la proposition du Gouvernement, nous ne sommes pas favorables à une transformation aussi radicale de l'AME ; seulement un migrant éligible sur deux y a recours, faute de connaissance du dispositif. Durcir les conditions d'accès et la couverture santé des migrants risque d'aggraver l'état de santé de cette population déjà précaire et de reporter la charge des soins sur les hôpitaux. Ainsi, selon l'issue des discussions, soit nous voterons en faveur de la mission, soit nous nous abstiendrons. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, année après année, la mission « Santé », composée des programmes 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », et 183, « Protection maladie », se résume toujours davantage à un débat centré sur l'aide médicale de l'État. Cette attention exacerbée portée à l'action n° 02 du programme 183 s'explique sans doute par le fait que l'AME absorbe progressivement la quasi-totalité de l'enveloppe dévolue à la mission « Santé », soit 82 % de celle-ci pour 2020, contre près de 45 % en 2010.

Pour 2020, les modifications de périmètre du programme 204 le conduisent à enregistrer une baisse de ses crédits de 58 %, alors que le budget de l'AME restera lui sensiblement inchangé par rapport à 2019. Cet automne, sur fond de débat sur la politique migratoire, l'aide médicale de l'État est la cible de nombreuses critiques et d'une réforme gouvernementale, alors même que le rapport de l'IGAS et de l'IGF d'octobre note que l'AME « n'est pas un outil de politique migratoire Concernant la gestion du dispositif, je souligne plusieurs évolutions intéressantes. Grâce notamment à une stabilisation du nombre de bénéficiaires, l'AME jouit d'une plus grande sincérité budgétaire.

Aussi, comme l'année dernière, je salue la position responsable et mesurée de notre rapporteure pour avis, Corinne Imbert. L'AME est une nécessité humanitaire, sanitaire et économique. À sa manière, elle participe à la politique publique de prévention sanitaire. Un droit de timbre et l'accès aux seuls soins d'urgence, comme le propose le rapporteur pour avis de la commission des finances, seraient tout bonnement contre-productifs. Les gains visés à court terme seraient dépassés par les coûts induits, notamment le recours aux urgences. Selon les référentiels des groupes politiques, l'AME incarne soit un mal nécessaire, soit le salut de notre nation. Cependant, en définitive, dans une vision purement pragmatique, l'AME est et restera une aide indispensable, avec un rapport bénéfices-risques avantageux. Est-il nécessaire de remettre en perspective le montant de l'AME face à celui de la consommation de soins et de biens médicaux en France ? J'en viens à la réforme proposée par le Gouvernement. une nouvelle fois le mauvais signal envoyé au Parlement par le Gouvernement, qui introduit sa réforme par voie d'amendements, la nuit même précédant l'examen de la mission « Santé » par l'Assemblée nationale. Certes, madame la secrétaire d'État, vous attendiez la remise du rapport de l'IGAS et de l'IGF pour agir. Mais celui-ci peine, en définitive, à trancher le débat et à apporter des éléments objectivables et chiffrés face aux nombreuses rumeurs et fantasmes. La mission La mission évoque des « suspicions de migrations pour soins » et rejette l'idée d'une réduction du panier de soins. Elle propose plutôt de conditionner la dispensation de certains soins à un délai d'ancienneté. À mon sens, les pistes les plus pertinentes de réforme de l'AME sont à chercher du côté de la simplification des échanges d'informations et des procédures entre les CPAM et les hôpitaux. Enfin, je rappelle le point de vigilance évoqué par Mme Imbert. Le conditionnement de l'accès à certains soins pour les bénéficiaires de l'AME devra pleinement laisser aux soignants une marge d'appréciation suffisante dans l'évaluation des besoins de chaque patient. le risque ? Décourager un recours aux soins, entraînant une explosion des dépenses de santé et des maladies infectieuses. Pour conclure, je m'interroge sur le devenir de la mission « Santé hors aide médicale de l'État. Ne faudrait-il pas la refonder, en s'appuyant sur quelques programmes forts ? C'est le sens de l'amendement que je défendrai avec mon collègue Jean-François Longeot. La maladie de Lyme est l'une des dix maladies infectieuses les plus fréquentes en France. Le diagnostic, la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique, laissant les malades dans une errance thérapeutique et dans un désert d'incertitude. La recherche est un acteur majeur de la prévention. Nous proposons donc de créer un programme spécifique « Recherche contre les maladies vectorielles à tiques », abondé à hauteur de 5 millions d'euros. mais elle constitue une première étape. C'est bien moins que les 15 millions d'euros d'économies demandées à l'AME. Je vous invite à répondre à cet appel des parlementaires, madame la secrétaire d'État. Le groupe Union Centriste votera les crédits de la mission « Santé », tels qu'ils ont été présentés à la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à la veille de la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est utile de rappeler que l'ensemble des crédits de la mission « Santé » ne représentent qu'une partie infime des moyens de notre politique publique en matière de santé. La dotation globale de cette mission s'élève, ainsi, à un peu plus d'un milliard d'euros en 2020, bien loin des 205 milliards de crédits consacrés aux dépenses de la seule branche de l'assurance maladie. Comme l'ont parfaitement expliqué nos collègues rapporteurs, Corinne Imbert et Alain Joyandet, dont je salue les travaux, les crédits de cette mission sont concentrés dans le programme 183, « Protection maladie », principalement consacré au financement de l'AME, qui représente 82 % des crédits de la mission. Par ailleurs, le financement des deux principaux opérateurs rattachés au programme 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », que sont l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Santé publique France, est transféré à partir de 2020 à l'assurance maladie. Certes, la simplification des circuits de financement des agences sanitaires est nécessaire. Toutefois, la succession des transferts a entraîné une diminution de 70 % des crédits versés à ce programme depuis 2012. Comme l'a fort justement souligné notre collègue Corinne Imbert, cette constante diminution des crédits dudit programme pose la question de la taille critique nécessaire au meilleur pilotage par l'État de la politique de santé publique. Plus largement, nous devons nous interroger sur le devenir de ce programme, et même sur celui de la mission « Santé ». J'en viens au programme 183, qui provoque, chaque année, des débats passionnés au sein de notre assemblée. Ce sujet mérite que nous l'abordions de manière sereine. Des mesures sur l'AME ont été présentées le 6 novembre dernier, à l'issue du comité interministériel sur l'immigration. Ces annonces ont conduit le Gouvernement à déposer des amendements, lors de l'examen en séance publique par les députés, de la mission « Santé », le 7 novembre dernier. Plusieurs mesures ont été adoptées visant à clarifier la condition de résidence et l'obligation de comparution physique devant les services. Pour les soins non vitaux, un délai d'ancienneté et un accord préalable ont été mis en place. Ces mesures ont conduit à une baisse de 15 millions d'euros de l'AME, ramenant son budget à 919 millions d'euros. Tout le monde dans cet hémicycle reconnaît qu'un dispositif d'accès aux soins d'urgence pour les étrangers, y compris en situation irrégulière, est tout à fait nécessaire, pour des raisons humanitaires et des raisons sanitaires évidentes. Toutefois, pour qu'un dispositif aussi indispensable puisse être défendu devant nos concitoyens, il faut qu'il soit mieux encadré. Quand le coût de l'AME augmente de 46 % entre 2011 et 2020, il est légitime de s'interroger sur les causes de cette évolution. Le Gouvernement estime que le renforcement de la lutte contre la fraude à l'AME permettra de limiter l'inflation de cette dépense en 2020. Si nous considérons qu'une telle démarche va dans le bon sens, nous pensons que ces effets seront insuffisants. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains, dans sa grande majorité, soutiendra la position du rapporteur spécial, M. Joyandet. La parole

Monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial, madame la rapporteure pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, vous étudiez aujourd'hui le budget de la mission « Santé » de la loi de finances pour 2020. Ce budget est marqué par une évolution importante de son périmètre, du fait du transfert à l'assurance maladie du financement de l'ANSM et de l'ANSP, d'où une baisse de 20 % des crédits de la mission. Ces crédits ne représentent toutefois qu'une petite partie des financements que les pouvoirs publics consacrent à la politique de santé. Ils sont, pour l'essentiel, discutés dans le cadre du PLFSS.

Cette dernière verra par ailleurs sa subvention augmenter de 8 millions d'euros, correspondant à la compensation de la suppression de la taxe sur le vapotage. Comme la ministre vous l'avait annoncé l'année dernière, nous avons poursuivi notre réflexion sur un financement intégral par l'assurance maladie de l'ANSM et de l'ANSP, ce qui nous amène à transférer le financement de ces deux opérateurs dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. L'activité de ces deux agences a en effet trait à des produits, les médicaments, ainsi qu'à une activité, la prévention, dont l'essentiel du financement dépend déjà de l'assurance maladie. Ce transfert renforce donc la cohérence des leviers d'action du ministère et n'altère en rien la possibilité pour l'État d'assumer ses responsabilités : la fonction de tutelle stratégique et de tutelle financière de ces deux agences reste inchangée. Les crédits de prévention au sein du programme 204 s'élèvent à 53 millions d'euros, après transfert de l'ANSP. Ce montant ne représente toutefois, je le rappelle, qu'une part très modeste du financement de la prévention. La création, cette année, d'un document de politique transversale permet ainsi de préciser que ces crédits représentent à peine plus de 1 % des presque 3 milliards d'euros qui seront consacrés en 2020 à la prévention sanitaire par le budget de l'État. la prévention dépasse très largement le champ de ce budget de l'État. Il faut en effet considérer l'ensemble des financements disponibles, quel qu'en soit le support, pour apprécier l'évolution des moyens consacrés à la prévention. Pour ne parler que de la prévention institutionnelle, elle est passée de 5,79 milliards d'euros en 2008 à 6,24 milliards d'euros en 2018, soit une augmentation de 7,8 %. Ces montants sont retracés dans l'annexe 7 au PLFSS. Pour autant, cette évolution n'est pas homogène sur les dix dernières années ; elle augmente de 0,3 % en moyenne par an entre 2008 et 2016, et de 2,7 % en moyenne par an entre 2016 et 2018. Cette tendance s'est accélérée en 2019, avec notamment l'élargissement des missions du fonds de lutte contre le tabac à la lutte contre les addictions, qui voit ainsi ses dépenses prévisionnelles s'élever à 119,7 millions d'euros en 2019, contre 100 millions en 2018 et 30 millions en 2017. Toutes les décisions qui ont été prises vont ainsi dans le sens d'une augmentation des crédits consacrés à la prévention. Les résultats sont probants. Grâce aux mesures phares relatives à la lutte contre le tabagisme du plan Priorité prévention, nous comptons 1,6 million de fumeurs quotidiens en moins entre 2016 et 2018. L'élargissement du document de politique transversale, pour le transformer en « jaune » budgétaire, me semble un apport intéressant des députés. Il faudra à l'avenir se poser la question de son articulation avec l'annexe 7 du PLFSS, pour éviter les doublons. Le programme 204 inclut également les dépenses d'indemnisation des victimes de la Dépakine. La gestion de ce dispositif d'indemnisation est, comme vous le savez, assurée par l'Oniam. Ce dispositif a connu une montée en charge progressive du fait de la complexité des questions juridiques et médicales soulevées lors de l'examen des dossiers. Elle va faire l'objet d'ajustements structurels visant à accélérer le traitement des dossiers. Le Gouvernement a déposé, lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, un amendement visant à simplifier le dispositif. À cet effet, les deux instances qui le composent, le collège d'experts et le comité d'indemnisation, vont être fusionnées. Par ailleurs, afin d'assurer une indemnisation plus facile des victimes, il est proposé de fixer dans la loi des dates à partir desquelles le lien entre le préjudice et le défaut d'information sera présumé : 1982 pour les malformations congénitales et 1984 pour les troubles du développement comportemental et cognitif. Les victimes pourraient ainsi être indemnisées plus aisément, sans voir leur dossier déclaré irrecevable. Enfin, à propos des crédits du programme 204, je veux signaler l'augmentation des moyens de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, sur laquelle repose exclusivement le système de santé pour l'ensemble de la population de ces deux territoires, et sa gratuité, au titre de la solidarité nationale. Sa dotation sera majorée en 2020 de 7 millions d'euros, pour la porter à 42,5 millions d'euros, afin également de développer en priorité la santé publique et la prévention, et de renforcer l'offre de soins, notamment grâce au déploiement de la télémédecine. Le deuxième programme de la mission, le programme 183, est consacré pour l'essentiel à l'AME. Le Gouvernement est attaché aux grands principes qui guident aujourd'hui notre politique d'accès aux soins et aux droits des personnes migrantes. Il n'est pas envisageable de les remettre en cause. Ce droit à la protection de la santé est un principe constitutionnel qui s'inscrit dans les engagements internationaux auxquels la France est partie. Ces dispositifs sont indispensables, non seulement pour des raisons humanitaires et de santé publique, mais aussi pour des raisons de maîtrise budgétaire. Nous savons que la prise en charge tardive d'une maladie est systématiquement plus coûteuse qu'une prise en charge précoce par la médecine de ville. Cependant, nous savons aussi que la dépense d'AME est dynamique : son montant est non négligeable, même s'il ne représente que 0,5 % des dépenses d'assurance maladie. maladie. La dépense d'AME alimente parfois une défiance, voire des fantasmes qu'il est difficile de déconstruire. Aussi, nous devons être responsables pour lutter contre les fraudes et les abus. C'est le sens des amendements adoptés, lors de l'examen à l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement. S'interroger sur l'efficience du dispositif, et l'amender en conséquence, c'est en garantir la pérennité. Mais nous devons aussi nous adapter aux problématiques particulières des migrants. Nous avons le devoir de bien prendre en charge les soins de ces personnes particulièrement vulnérables. Pour cela, nous devons poursuivre les démarches pour « aller vers » ces populations et les faire accéder aux soins ou aux droits. Dans le texte qui vous est aujourd'hui soumis, nous prévoyons ainsi de clarifier le droit applicable, en indiquant qu'il est nécessaire d'être depuis trois mois en situation irrégulière pour bénéficier de l'AME. Cela ne changera rien pour les personnes entrées en France de façon irrégulière, mais aura une incidence pour les détenteurs d'un visa de tourisme, car le délai de trois mois, qui leur est déjà applicable, commencera désormais à l'expiration de leur visa. de renforcer le contrôle de la résidence en France. Les demandes d'AME devront être déposées par les intéressés, en personne, dans une CPAM ou, par dérogation, par l'intermédiaire de l'hôpital ou d'une permanence d'accès aux soins de santé. L'objectif est d'éviter les demandes frauduleuses, transmises par courrier, de personnes qui ne se trouvent pas sur le territoire français. De plus, nous prévoyons de mettre en place une procédure d'accord préalable, pour certains soins programmés et non urgents. d'introduire un délai de carence de trois mois pour l'accès à la PUMa des demandeurs d'asile. Actuellement, les demandeurs d'asile bénéficient de règles dérogatoires, plus favorables que les dispositions appliquées aux autres assurés. Les demandeurs d'asile auront accès aux soins urgents pendant ce délai de trois mois. Seront notamment concernés les soins hospitaliers vitaux, le traitement des maladies infectieuses et les soins délivrés aux femmes enceintes et aux nouveau-nés.

contrairement à ce que vous affirmez, les mesures que vous présentez se traduiraient par une dégradation de la santé des personnes concernées, par un engorgement des services d'urgences et par une augmentation du coût total des soins dispensés.

en santé par titulaire de l'AME est inférieure à la dépense moyenne d'un assuré social. Certes, cette dépense a progressé.

Comme la protection universelle, l'aide médicale de l'État répond à des objectifs humanitaires et de santé publique, en permettant la prise en charge de mesures de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. Conformément aux engagements de maîtrise des dépenses publiques et de lutte contre les fraudes, nous souhaitons renforcer les contrôles. Ces derniers porteront sur les conditions d'éligibilité à l'AME, comme la durée du séjour et les ressources effectives des demandeurs. Ils pourront également avoir lieu, avoir lieu, en particulier pour les bénéficiaires qui ont le plus recours aux soins. Par ailleurs, le regroupement des demandes d'AME dans trois caisses primaires d'assurance maladie permettra un meilleur contrôle. loin de suivre un raisonnement purement budgétaire, nous avons refusé de remettre en cause le panier de soins. Nous ne souhaitons pas non plus réintroduire la participation financière des personnes admises. En effet, dans leur rapport

des reports de soins de la part de personnes dont l'état de santé était souvent dégradé. Il en est résulté un déport vers des soins hospitaliers plus coûteux, notamment du fait d'une prise en charge tardive. Monsieur le rapporteur

sociale et des familles, alinéa 5, après le mot « concerne », les mots « au titre des soins urgents, des risques sanitaires et épidémiologiques ».

préserver les dispositions de l'article L. 251-3, lequel précise que les modalités d'application de l'ensemble du chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État.

CRCE. Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

de l'AME, à des programmes de santé publique qui s'adressent à l'ensemble de la population. Pour cette seule raison, nous ne voterons pas ces amendements,

en 2017 puis à 67 000 nouveaux cas dénombrés par Santé publique France en 2018. C'est considérable : la maladie de Lyme fait désormais partie des dix maladies infectieuses les plus fréquentes en France. Nous avons tous été contactés pour différents cas. En l'absence de système de déclaration obligatoire organisé à grande échelle et compte tenu de l'insuffisante sensibilisation des médecins traitants au dépistage de cette maladie complexe, le recensement du nombre de cas avérés reste incomplet, sujet à extrapolation et, probablement, sous-évalué. Le diagnostic, la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique, laissant les malades dans une errance thérapeutique. Or, en l'absence de diagnostic rapide, les complications peuvent être lourdes et mener à des dommages irréversibles, chez les adultes, mais aussi, on le constate de plus en plus, chez les enfants. Sans nous prononcer sur ce que devrait être le diagnostic ou la prise en charge de la borréliose de Lyme, nous ne pouvons rester indifférents aux dizaines de témoignages de patients que nous recevons chaque année et qui font état de leur souffrance face à la maladie et à un parcours de soins particulièrement chaotique. Si le Gouvernement reconnaît le sérieux de la situation, il se refuse à augmenter l'effort indispensable de recherche sur ce thème. En apportant des crédits importants à la recherche fondamentale et appliquée sur cette maladie, cet amendement vise à améliorer durablement la vie des patients. Il est donc proposé de créer un programme spécifique « Recherche contre les maladies vectorielles à tiques », abondé à hauteur de 5 millions d'euros prélevés sur l'action n° 11, Pilotage de la politique de santé publique, du programme 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

et du financement. Le ministère de la santé travaille en lien étroit avec le ministère de la recherche, avec les agences sanitaires et d'autres organismes de recherche qui vont augmenter leur contribution aux projets consacrés aux maladies vectorielles.

véritablement des process d'innovation qui ne sont pas suffisamment reconnus. Nous savons que notre système ne reconnaît pas suffisamment les innovations, lorsqu'il n'y a pas de « comparateurs

est une maladie héréditaire qui touche l'hémoglobine. Cette protéine est essentielle à la fonction respiratoire. C'est elle qui permet le transport de l'oxygène dans notre organisme. Elle participe aussi à l'élimination aussi à l'élimination du dioxyde de carbone. Une telle maladie génétique est très répandue dans le monde. Apparue indépendamment en Afrique et en Inde, elle touche tout particulièrement les populations de ces régions. Mais les mouvements de populations l'ont rendue très présente en Amérique, tout particulièrement aux Antilles et au Brésil, et en Europe de l'Ouest. Cette pathologie touche plus de 20 000 malades en France et plus de 150 000 porteurs sains avérés. En France, 441 enfants drépanocytaires ont vu le jour en 2013, soit une prévalence d'un enfant atteint pour 1 900 naissances. Cela en fait la maladie génétique la plus fréquente en France. Toutefois, la prévalence est beaucoup plus importante dans les départements d'outre-mer et en région parisienne, où se concentrent les populations à risque. Aujourd'hui, personne ne connaît exactement le coût de la drépanocytose en France. On sait tout juste que le professeur Frédéric Galacteros, spécialiste de la drépanocytose, a présenté une étude américaine chiffrant à 1 million de dollars le coût d'un patient drépanocytaire- dans leur système de santé, c'est le coût total d'une vie de malade. Ce coût, assurément élevé, plaide en faveur d'une vraie politique de prévention et d'investissements dans la recherche de traitements moins onéreux. Beaucoup d'efforts sont à faire pour que le combat contre la drépanocytose rejoigne le niveau de ce qui existe pour les autres maladies génétiques. Cela suppose d'abord une information large auprès du corps médical, des paramédicaux, des laboratoires d'analyses- chacun peut contribuer à son échelle à la formation à ces problèmes -, des communautés concernées et du public en général, par l'intermédiaire de l'école et des médias. Mais rien ne pourra se faire sans recherche à tous les niveaux. Cet amendement vise donc à créer un programme spécifique intitulé « Recherche contre la drépanocytose » qui serait abondé à hauteur de 5 millions d'euros, prélevés sur l'action n° 11, Pilotage de la politique de santé publique, du programme 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

entre soins et recherche doit être particulièrement étroit. C'est pourquoi des efforts financiers importants sont réalisés pour soutenir des actions pour la recherche. Ainsi, le troisième plan national Maladies rares, lancé voilà un an, est doté d'un budget de près de 780 millions d'euros. Pour la filière de santé relative à la drépanocytose, la coordination des acteurs nationaux du programme européen de recherche sur les maladies rares est un enjeu majeur. Elle s'inscrit dans le programme prioritaire de recherche sur les maladies rares coordonné par l'Inserm. Ce travail déjà entamé cette année a défini les contours d'appels à projets destinés à la recherche sur les maladies rares, dont les patients atteints de drépanocytose pourront bénéficier. Des financements spécifiques de plus de 40 millions d'euros sont déjà prévus jusqu'en 2022.

Un dispositif de pharmacovigilance piloté par l'Anses a été mis en place dès 2014 pour surveiller les éventuels effets indésirables. Le Gouvernement a aussi engagé des actions pour réduire l'utilisation des pesticides des pesticides de 25 % d'ici à 2020 et de 50 % d'ici à 2025. Des mesures de protection des publics sensibles ont été adoptées. Les sources de financements prévues par le Gouvernement apparaissent suffisantes pour couvrir les besoins du fonds. L'avis est donc défavorable.

des crédits de la mission

car les personnes étrangères continueront d'être malades, un non-sens économique, car elles retarderont leurs soins et les symptômes s'aggraveront et nécessiteront des interventions plus complexes et plus longues, et enfin un non-sens humanitaire, car vous cédez aux fantasmes de la droite la plus extrême : plutôt que de maintenir des conditions d'accueil dignes de notre pays, vous les restreignez. Le professeur Frédéric Adnet, chef des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, qui

dernier : « Non. C'est un fantasme complet ! Je n'ai jamais observé et on ne m'a jamais rapporté de patients qui présenteraient leur carte d'AME pour faire soigner leur cancer. Je mets quiconque au défi de prouver l'existence d'un tel tourisme médical. Il n'existe aucun chiffre, seulement des bruits de couloir. Les patients bénéficiaires de l'AME n'ont pas calculé de venir en France pour soigner des pathologies chroniques. Pourtant, je travaille dans l'hôpital le plus proche de l'aéroport de Roissy, donc si le tourisme médical existait, on le verrait chez nous. » Il conclut par ces mots : « L'AME a donc un effet de médecine préventive et permet d'éviter la dissémination des pathologies contagieuses. [ ...] On a tout intérêt, au contraire, à maintenir ce dispositif et même à l'étendre aux personnes qui résident depuis moins de trois mois sur le sol français. » Tout est dit, mes chers collègues. C'est pour cette raison que nous soutenons totalement l'amendement de nos collègues socialistes.

Parce que, on l'a dit, les démarches sont trop compliquées et que l'ignorance de l'existence même de ce dispositif pèse sur ces personnes. Tel est le résultat d'une étude réalisée par l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé et l'université de Bordeaux, qui permet pour la première fois de mieux dessiner le profil des bénéficiaires de l'AME. En réalité, seul un migrant en situation irrégulière sur deux, pourtant éligible à l'aide médicale de l'État, y a recours.

Dans l'ensemble, si le non-recours à l'AME reste fréquent, c'est que 33 % déclarent n'avoir jamais entendu parler de ce dispositif, et 41 % ont abandonné les démarches qui sont trop compliquées. Cela a déjà dit dans nos débats, mais je je m'appuie là sur une étude. Je sais que plusieurs de mes collègues sont friands de statistiques : eh bien, en voilà ! Finalement, toutes les complexités administratives qui ont été mises en place par les gouvernements successifs

Quel est l'avis du Gouvernement ? Les « jaunes » et les « oranges » budgétaires, aussi appelés documents de politique transversale, ont tous deux vocation à retracer l'effort financier global dédié à une politique interministérielle.

est dotée de 25,5 milliards d'euros de crédits de paiement en 2020. Ces crédits progressent ainsi de 6,7 % par rapport à 2018, soit une augmentation de près de 1,6 milliard d'euros. Cette hausse significative est principalement due au dynamisme structurel et aux revalorisations de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), dont les dépenses sont estimées à 20 milliards d'euros pour 2020. Malgré cette hausse des crédits et les revalorisations que nous saluons, ce budget n'est pourtant pas pleinement satisfaisant, madame la secrétaire d'État. D'abord, ce budget intègre, comme les années précédentes, de discrets « coups de rabots » touchant les plus fragiles revalorisation à 0,3 % en 2020 de la prime d'activité et de l'AAH ; baisse de l'abattement portant sur les revenus d'activité pris en compte dans le calcul de la prime d'activité ; suppression du complément de ressources pour les bénéficiaires de l'AAH notamment. Ensuite, ce budget est entouré d'un certain nombre d'incertitudes, qui nous inquiètent. En premier lieu, la montée en charge extrêmement dynamique des dépenses de prime d'activité qui a occasionné des difficultés de gestion dans les caisses d'allocations familiales (CAF), comme nous avons pu le constater lors de nos déplacements dans les CAF du Nord et du Val-d'Oise. Les CAF ont reçu, du 1 janvier au 30 avril 2019, plus de 1,4 million de demandes, contre 276 000 à la même période en 2018. Le nombre de foyers allocataires de la prime d'activité a ainsi augmenté de 47 % entre septembre 2018 et mars 2019, pour atteindre aujourd'hui 4,1 millions de foyers bénéficiaires. Outre le nombre de bénéficiaires, l'évolution de leur profil nous amène à nous interroger. D'après un rapport du Gouvernement remis au Parlement, ce sont les tranches de revenus les plus élevés qui progressent parmi les bénéficiaires.

Le Gouvernement semble avoir fixé deux lignes rouges, sur lesquelles je serai extrêmement vigilant : premièrement, aucune conditionnalité en termes d'activité ne sera exigée pour le versement du revenu minimum s'agissant du handicap deuxièmement, les moyens mobilisés aujourd'hui pour le handicap devront lui rester affectés. Par ailleurs, outre son périmètre, des incertitudes entourent le financement

Dernier sujet d'inquiétude que je souhaitais aborder et qui concerne d'ailleurs également les départements : le financement de l'accueil des mineurs non accompagnés (MNA), dont l'enveloppe prévue n'est toujours pas à la hauteur des enjeux. L'ADF estime aujourd'hui à 2 milliards d'euros le coût induit par l'évaluation et la prise en charge de ces mineurs, quand le budget de l'État atteint péniblement les 162 millions d'euros. Pourquoi, madame la secrétaire d'État, l'État, qui s'y était d'ailleurs engagé, ne reprend-il pas à sa charge une partie du dispositif, qui devrait légitimement lui revenir au titre de ses missions régaliennes ? M. le Premier ministre l'avait d'ailleurs annoncé quand il a rencontré en 2017 les départements de France lors de leur congrès annuel. Malgré ces insuffisances que je regrette vivement et au vu de la hausse des crédits,

par la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, lancée par le Gouvernement en octobre dernier. Si l'ambition de ce plan est louable, nous nous interrogeons sur son financement et ses modalités de mise en oeuvre.

Autre sujet d'inquiétude, le financement de l'aide alimentaire, qui fut l'objet de notre précédent rapport de contrôle. Le système d'aide alimentaire français, qui bénéficie aujourd'hui à près de 5,5 millions de personnes, apparaît plus que jamais fragilisé par les difficultés de gestion liées au Fonds européen d'aide aux plus démunis. Ces difficultés font peser de vrais risques budgétaires pour la France : au bas mot, 70 millions d'euros dus à des non-remboursements de la part de la Commission européenne devraient être compensés sur le budget de l'État. C'est assez dramatique, d'autant que la prochaine programmation se profile. Madame la secrétaire d'État, je sais que vous suivez ce dossier de près, mais il est impératif que l'État tire les conséquences de ces défaillances, pour que,, les bénéficiaires, les plus fragiles de nos concitoyens, ne soient pas encore les victimes collatérales de sa mauvaise gestion. Par Par ailleurs, sur ce sujet de l'aide alimentaire, je souhaitais vous interroger, madame la secrétaire d'État, sur l'incohérence de la réforme du mécénat que vous mettez en oeuvre. Les associations d'aide alimentaire dites « loi Coluche » ont été exclues du champ d'application du dispositif. Néanmoins, cette dérogation s'applique seulement aux structures « qui procèdent à la fourniture gratuite de repas », et tend donc à exclure les épiceries solidaires, dont le modèle reposant sur la participation symbolique des bénéficiaires pourrait être remis en cause, ce qui serait très regrettable.

Plus que jamais, cette priorité politique, déclarée comme telle par le Gouvernement, doit faire l'objet d'un passage des paroles aux actes. Habitué à s'attribuer la création de mesures déjà existantes ou à faire fi des politiques passées, le Gouvernement semble, sur ce sujet, se heurter à l'épineuse question budgétaire. Nous souhaitons ainsi faire trois séries d'observations pour rétablir la réalité des chiffres. Tout d'abord, nous sommes très loin du milliard d'euros annoncé pour l'égalité et la lutte contre les violences faites aux femmes, comme nous avons pu le démontrer dans notre rapport. Nous constatons même la diminution des crédits consacrés à la lutte contre les violences, au sein du programme 137, entre 2019 et 2020. Par ailleurs, aucune mesure budgétaire concrète n'a été annoncée pour financer les mesures du Grenelle contre les violences conjugales. Interrogé, le cabinet de Mme Schiappa n'a, semble-t-il, pas jugé utile de nous répondre. Madame la secrétaire d'État, pourriez-vous peut-être nous éclairer sur la budgétisation de ces mesures annoncées ? Enfin, les associations ont dû affronter une hausse sans précédent de demandes depuis le mouvement #MeToo, sans bénéficier parallèlement, pour certaines d'entre elles, de hausse de crédits. Par ailleurs, le peu de considération du ministère pour les associations nous laisse quelque peu perplexes : certaines structures n'ont pas encore reçu leur subvention au titre de 2019 ni d'informations quant au renouvellement de leur convention pluriannuelle débutant en 2020.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens d'abord à saluer l'effort budgétaire important qui a été consenti en faveur de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis 2018, bien que celle-ci reste inférieure au seuil de pauvreté. Toutefois, l'augmentation de 0,3 % proposée pour 2020 afin de freiner la hausse des dépenses aura pour effet de dégrader dès l'an prochain le pouvoir d'achat des allocataires. Nous devrons veiller à ce que cette sous-revalorisation n'amorce pas un nouveau décrochage. L'AAH, parce qu'elle s'adresse à des personnes confrontées aux plus grandes difficultés, voire à l'impossibilité de s'insérer ou de se maintenir dans l'emploi, ne devrait pas être considérée comme un minimum social de droit commun. À cet égard, la baisse du plafond de ressources applicable aux allocataires en couple entre 2018 et 2019 a sans doute été trop brutale et a contribué, avec la suppression du complément de ressources, à la perception mitigée de leur situation par les bénéficiaires de l'AAH. Pour les mêmes raisons, je suis profondément réservé à l'égard d'une absorption de l'AAH dans un revenu universel d'activité. L'exercice d'harmonisation des bases de ressources a ses limites, s'agissant d'une allocation conçue au fil du temps pour répondre aux besoins d'un public bien particulier. En revanche, l'idée d'un rapprochement avec l'allocation supplémentaire d'invalidité est intéressante et permettra de simplifier le parcours des allocataires. La commission propose de préciser par coordination son mode de calcul. S'agissant de la prime d'activité, la revalorisation exceptionnelle du « bonus » individuel au 1 janvier 2019 semble avoir réconcilié ses objectifs de soutien du pouvoir d'achat des familles aux revenus modestes et d'incitation à l'exercice d'une activité professionnelle, au prix d'un effort financier considérable, et assurément sous-estimé pour 2020. Toutefois, après quatre ans d'existence de la prime, son impact réel sur l'emploi reste impossible à quantifier. Sur ce point, il semble que le Gouvernement continue de considérer le taux de recours et l'augmentation des dépenses comme des objectifs en soi, sans s'interroger plus avant sur les effets complexes de cette prestation. Elle aura du moins le mérite de réduire, en 2019, un taux de pauvreté qui a bondi en 2018 de 14,1 % à 14,7 %, selon les données provisoires publiées par l'Insee. Quant à la stratégie Pauvreté, la volonté d'établir un rapport de confiance avec les acteurs territoriaux doit être relevée. Toutefois, plusieurs départements ont vu leurs relations avec l'État se durcir depuis le début du processus de contractualisation, et les collectivités s'inquiètent de voir cette méthode se traduire par une nouvelle forme de tutelle de l'État. Au sein du budget de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui reste stable à l'euro près en dépit des ambitions affichées, la commission estime que le la commission estime que le financement de la lutte contre la prostitution devrait être maintenu à son niveau de 2019. Enfin, la commission propose, cette année encore, un amendement symbolique, mais ô combien important, qui vise à créer au sein de la mission un nouveau programme budgétaire consacré à l'évaluation et à l'hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés, afin que soit officiellement reconnue la compétence de l'État en cette matière. Sous ces réserves, la commission a donné un avis favorable aux crédits de la mission. Mes chers collègues, je vous de la mission. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes

mes chers collègues, cette mission porte un magnifique titre, « Solidarité, insertion et égalité des chances », qui laisse miroiter des ambitions d'harmonie, de cohésion sociale et d'attention aux personnes les plus fragiles. Il y a de quoi faire Le nombre de pauvres a augmenté et la pauvreté touche désormais plus de 9 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants- on peut hélas ! deviner le destin qui leur est promis. Sept cents enfants à la rue sont recensés à Paris. Les 10 % les plus pauvres voient leur pouvoir d'achat régresser. Une famille sur deux déclare ne pouvoir financer le logement étudiant de son enfant. Les inégalités se creusent. Quant aux revenus et aux fortunes des plus riches, ils s'envolent à une hauteur « sans précédent », selon la formule que vous employez à l'envi pour la moindre petite chose. femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint et 22 000 femmes subissent des violences physiques ou sexuelles. La France est championne du monde du déterminisme social. Ainsi, les enfants pauvres d'aujourd'hui seront les adultes pauvres et révoltés de demain, et la violence ne cessera d'augmenter. « Vaste programme », aurait dit, sur un autre sujet le général de Gaulle. Vaste programme, qui justifiait, en matière de solidarité et d'égalité des chances, une forte détermination.

En réalité, votre politique sur cette mission se situe dans le droit fil de toutes les autres, marquée par les déclarations triomphalistes que la maigreur des efforts et des effets est loin de justifier, et par des présentations en trompe-l'oeil qui n'abusent plus personne, tant la parole du Gouvernement est décrédibilisée. Ainsi en est-il de l'affirmation d'un gain de pouvoir d'achat de 100 euros par la prime d'activité. La vérité exige de déduire l'augmentation normale du SMIC et la perte liée à l'inflation. Il en est ainsi, encore, du milliard d'euros annoncé par Mme la ministre, une annonce qui relève pour le moins d'une présentation largement enjolivée de la réalité. Ce gouvernement manifeste une affection singulière pour les primes, au détriment des augmentations de salaire : prime d'activité quand une augmentation de salaire était attendue, prime pour les agents hospitaliers qui ne s'en satisfont pas ... Il est vrai que la prime engage beaucoup moins. Ainsi pouvez-vous pratiquer sur les allocations diverses et les primes une désindexation qui réduira le pouvoir d'achat de celles-ci de près de 1 %. Pourquoi cet acharnement à faire payer les plus fragiles ? Il est vrai qu'ils ont moins de moyens pour manifester leur mécontentement, sauf par la violence accrue ou l'espoir vain et dangereux du recours aux extrêmes. Ils sont les malheureuses victimes de vos politiques. Près de 1,2 million de chômeurs chômeurs et leur famille vont progressivement sombrer dans le dénuement le plus tragique. Ils viendront augmenter la cohorte croissante des personnes pauvres. La baisse des aides personnalisées au

Les salariés aux revenus inférieurs à la moitié du SMIC sont écartés du bénéfice de la prime d'activité, de même que les étudiants qui, de surcroît, pour certains, subiront douloureusement les nouvelles références en matière d'APL. Certes, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés apprécieront l'augmentation, même atténuée par la désindexation, de 860 à 900 euros de leur allocation. Mais n'est-il pas mesquin de l'assortir de la suppression du complément de ressources, qui pouvait atteindre 170 euros et garantissait un minimum de revenus à ceux que le handicap empêche de disposer d'un salaire ? N'est-ce pas petit et injuste de plafonner l'AAH d'un couple en l'affectant d'un coefficient de 1,81, alors qu'il était de 2, soit une perte de 10 % des revenus ? Cette mesure pénalisera Riche et bien portant, on est l'objet de beaucoup de sollicitude. Pour les autres, ça va être dur ... Pourtant, un PLF devrait être un moment de créativité, d'enthousiasme, d'innovation pour améliorer sans cesse les conditions du vivre ensemble. Comment tirer quelque enthousiasme d'une proposition inodore et sans saveur ? L'examen de quelques aspects de votre politique est édifiant. En matière de lutte contre la pauvreté, on passe certes de 150 millions à 215 millions mais pour plus de 9 millions de pauvres ... Dérisoire ! Totalement dérisoire ! Il est vrai que l'essentiel sera apporté par les départements, qui auraient mauvaise presse auprès de leurs habitants s'ils refusaient de s'y engager. et les hommes, il n'y a pas 1 milliard d'euros, contrairement aux grandiloquentes déclarations, mais seulement 557 millions d'euros, dont une bonne partie pour des actions internationales. La seule prise en charge des femmes victimes de violences conjugales nécessiterait entre 500 millions et 1 milliard d'euros, selon le Haut Conseil à l'égalité, dont vous déciderez peut-être avez décidé celle de l'Observatoire de la pauvreté. Plus de thermomètre, plus de malade ... Pour l'heure, l'inscription budgétaire est limitée à 280 millions d'euros. Le reste est littérature Pourtant, les annonces furent solennelles et les mots forts. Les termes « électrochoc », « changement de paradigme » cherchent à masquer, mais cachent mal les insuffisances. Il n'y a pas un sou supplémentaire. Les actions de prévention propres à éviter de nouvelles victimes ne sont que des reprises. Les Françaises et les Français qui manifestaient en grand nombre

anciens migrants et les moyens affectés à l'accompagnement des femmes en sortie de prostitution sont en nouvelle décroissance, loin des déclarations sur la volonté de les aider à sortir de l'enfer.

Détruire la misère ! Oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. le devoir n'est pas rempli. » Aussi, je me félicite que le budget pour 2020 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » augmente de 6,7 % par rapport à 2019. Cela représente en effet près de 1,6 milliard d'euros de crédits supplémentaires et un total de 25,5 milliards d'euros en faveur des plus vulnérables et des plus démunis. hausse est essentiellement due à l'augmentation exponentielle des dépenses de prime d'activité et d'allocation aux adultes handicapés, qui figurent parmi les trois principales dépenses sociales financées par la mission, avec les mesures de protection juridique des majeurs. Elles représentent à elles seules plus de 80 % des crédits de la mission en 2020, soit 20,7 milliards d'euros. La prime d'activité et l'AAH constituent des acquis sociaux à pérenniser. Aussi, je ne peux que saluer l'augmentation du budget qui leur est alloué. Pour autant, à l'instar des rapporteurs spéciaux, je regrette que cette hausse s'accompagne « de discrets coups de rabot touchant les plus fragiles la protection juridique des majeurs est en hausse. Les crédits alloués à cette action s'élèvent à 688,4 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 3 % par rapport à 2019 due à l'augmentation continue du nombre de mesures. Ces crédits financent près de 497 000 mesures de protection- tutelles, curatelles ou sauvegardes de justice -, contre 484 656 en 2019, confiées à des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ils financent également l'information et le soutien aux tuteurs familiaux. On compte aujourd'hui 730 000 majeurs protégés, et ce nombre est voué à augmenter chaque année, car il existe de nombreux territoires- je pense particulièrement à Saint-Martin -où toutes les familles n'ont pas pris l'habitude de saisir le juge des tutelles. Il est donc indispensable de flécher des crédits sur l'information aux familles, tout en ayant conscience que cela augmentera mécaniquement le nombre de majeurs protégés et donc le volume de crédits engagés par l'État. En dehors de ces trois grandes dépenses sociales, la mission en intègre d'autres, tout aussi importantes. Je pense bien sûr à la nouvelle stratégie interministérielle de lutte contre la pauvreté. Récemment, l'Insee fixait le taux de pauvreté pour 2018 à 14,7 % de la population, soit une hausse de 0,6 point par rapport à 2017. Cela porte à 9,3 millions le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Aussi, je salue la montée en charge de cette mission, qui s'appuie sur une approche contractuelle avec les départements, véritables chefs de file en matière d'action sociale dans les territoires. Par ailleurs, des mesures d'investissement social- petits-déjeuners gratuits à l'école, tarification sociale pour l'accès à la cantine, déploiement des points-conseil budget, etc. -continuent à être financées à hauteur de 44 millions d'euros. Autre dispositif vital, l'aide alimentaire, qui a bénéficié à 5,5 millions de personnes en 2017. Alors que s'est ouverte, il y a trois jours, la trente-cinquième campagne d'hiver des Restos du coeur, je souhaiterais rendre hommage à l'ensemble des associations et des bénévoles qui oeuvrent quotidiennement auprès des plus démunis. L'aide alimentaire offre une aide d'urgence, mais représente surtout le point de contact privilégié pour permettre un accompagnement vers l'autonomie. Les crédits de l'action sociale s'élèvent à 74,5 millions d'euros, dont plus de la moitié- 40 millions d'euros -sont consacrés à la contribution de la France au Fonds européen d'aide aux plus démunis en complément de la contribution de l'Union européenne, qui s'élève à 75,6 millions d'euros. Je souscris toutefois aux inquiétudes exprimées par les rapporteurs spéciaux sur la fragilisation du système d'aide alimentaire français en raison des difficultés de gestion liées au FEAD, qui font peser des risques de pertes budgétaires importantes sur la France. Pour le reste, je relève, comme les rapporteurs, plusieurs points d'incertitude la montée en charge particulièrement dynamique des dépenses de prime d'activité, qui a occasionné des difficultés de gestion dans les CAF, la mise en oeuvre du revenu universel d'activité, dont le périmètre et le financement ou encore la diminution des crédits affectés à la prévention des violences faites aux femmes. S'agissant de ce dernier point, je m'interroge sur cette baisse, alors que 131 femmes ont été tuées en France depuis le début de l'année par leurs compagnons ou ex- compagnons.

de crédits supplémentaires, même s'il faut tenir compte, entre-temps, des crédits ouverts dans le projet de loi de finances rectificative pour 2019, à hauteur de 839 millions

Notons que les quatre programmes qui composent la mission sont en augmentation, pour s'établir à 11,9 milliards d'euros pour le programme 304, « Inclusion sociale et protection des personnes », 12,2 milliards d'euros pour le programme 157, « Handicap et dépendance », 30 millions d'euros pour le programme 137,

mais également la montée en puissance de la stratégie interministérielle de lutte contre la pauvreté, dont une partie des actions relève du programme 304, notamment la lutte contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou les maraudes mixtes entre les pouvoirs publics et les acteurs associatifs. Attardons-nous Attardons-nous dans un premier temps sur la prime d'activité. Comme chacun le sait, celle-ci a été sensiblement revalorisée en décembre dernier pour répondre à la mobilisation des « gilets jaunes », à hauteur de 90 euros au niveau du SMIC.

En un an, le nombre d'allocataires a ainsi augmenté de 47 %, soit près de 1,25 million de nouveaux bénéficiaires de la prime de septembre 2018 à mars 2019. La réforme a permis d'augmenter les montants moyens de prime d'activité versés, et en même temps

La mission inclut aussi les crédits du programme 137, « Égalité entre les femmes et les hommes », érigée « grande cause du quinquennat » par le Président de la République. L'égalité entre les femmes et les hommes est appuyée dans ce programme, entre autres, par des actions d'accompagnement et de prise en charge des victimes de violences physiques et sexuelles, de prévention et de lutte contre la prostitution et la traite humaine ou encore de soutien à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. En raison de l'importance de ces sujets, nous ne pouvons que nous réjouir de la « sanctuarisation » de ces crédits. Avant de conclure, en s'appuyant sur le rapport de leur collègue Patricia Schillinger,

Enfin, malgré toutes les augmentations précédemment citées, la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » fait l'effort de participer à la baisse du déficit public,

nous discutons ce soir des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », dans le cadre du projet de loi de finances. La solidarité, « la grande chose de la démocratie », pour reprendre le mot de Victor Hugo, occupe chaque année une place singulière dans les discussions budgétaires. C'est moins à cause des crédits qui lui sont consacrés, même s'ils sont importants, avec près de 25 milliards d'euros pour 2020, que parce qu'elle se trouve au fondement du modèle social français et règle les modalités du vivre ensemble. Rien d'étonnant, donc, à ce que les crédits excèdent finalement ceux qui avaient été fixés initialement, car la solidarité se laisse mal encadrer par des prévisions trop rigides. Ainsi, à périmètre constant, les crédits de la mission ont progressé de 6,7 % entre 2019 et 2020, soit une augmentation de 1,6 milliard d'euros. Ces crédits ont largement dépassé le plafond de dépense triennal fixé par la loi de programmation 2018-2022 à 22 milliards d'euros. Le budget consacré à cette mission est aussi porté par des dépenses fiscales dynamiques, qui ont augmenté de 20 % au cours des dix dernières années. Je pense notamment à l'abattement sur les pensions et au crédit d'impôt sur le revenu pour frais de garde. Ces dépenses fiscales poursuivent des objectifs louables. Elles soutiennent des politiques qui sont appréciées par nos concitoyens, car elles sont utiles pour la société. Mais les dépenses fiscales ne sont pas les seules dépenses dynamiques de la mission. Certaines dépenses se caractérisent même par un dynamisme structurel elles sont donc amenées à augmenter « par construction », et ce serait en écorner le principe que de chercher à en diminuer le montant. C'est tout particulièrement le cas de l'allocation aux adultes handicapés, qui représente environ 40 % des crédits et plus de 10 milliards d'euros. Le vieillissement de la population et le recul de l'âge de départ à la retraite, d'une part, et le faible taux de sortie des allocataires de cette allocation, d'autre part, constituent deux facteurs qui orientent le montant de cette allocation à la hausse. Je salue la décision du Gouvernement d'en revaloriser le montant à taux plein à hauteur de 900 euros. Cette dépense de solidarité fait honneur à notre société et son augmentation nous oblige. toutes les dépenses intégrées dans la mission ne sont pas structurelles. D'autres sont plus conjoncturelles, mais non moins importantes en termes de montants. C'est le cas de la prime d'activité, qui devrait représenter, en 2020, près de 10 milliards d'euros et concerner un actif sur quatre. Les mesures annoncées par le Président de la République il y a un an y ont largement contribué. Le Sénat les a acceptées comme des mesures d'urgence, en faisant preuve de responsabilité, mais nous pouvons désormais nous interroger sur leur cohérence à long terme avec le projet politique du Gouvernement. La hausse de la prime d'activité est emblématique de l'incertitude qui plane sans cesse au-dessus de cette mission : c'est sur elle que sont imputées les mesures onéreuses destinées à endiguer les colères populaires. Pour ainsi dire, l'instabilité y fait figure de constante ... Pourtant, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des sommes engagées. Cette incertitude pèse avant tout sur le budget de l'État. On l'a vu avec les mesures votées au coeur de la crise, en décembre 2018. On le pressent avec le futur revenu universel d'activité annoncé pour 2020 par le Président de la République. En effet, on ignore pour le moment la mécanique de ce dispositif, si bien qu'il semble impossible d'évaluer aujourd'hui le coût de cette mesure qui devrait pourtant voir le jour demain. Je partage les deux interrogations soulevées par les rapporteurs spéciaux : l'AAH sera-t-elle absorbée par le dispositif ? Quel rôle pour les départements dans ce futur pilier des politiques de solidarité ? L'incertitude pèse également sur les collectivités territoriales, madame la secrétaire d'État, singulièrement sur les départements qui traduisent notre modèle social sur le terrain. au rôle des départements dans le futur, le sujet très sensible du financement des mineurs non accompagnés les préoccupe déjà grandement, et à raison. En effet, la hausse de 20 % des crédits qui y sont consacrés apparaît en décalage avec la réalité du terrain. France (ADF), il faudrait mobiliser au moins 2 milliards d'euros pour accueillir les quelque 32 000 individus concernés. Les départements sont en première ligne et ils craignent que l'État ne se décharge sur eux. Nous espérons, madame la secrétaire d'État, que vous pourrez les rassurer à ce sujet, et nous avec. Enfin, le groupe Les Indépendants se réjouit que le Gouvernement ait prévu de faire participer le ministère des solidarités et de la santé aux efforts de réduction de la dépense publique, notamment pour ce qui concerne la rationalisation des effectifs et de l'immobilier. Vous l'aurez compris, notre groupe partage l'esprit d'une politique de solidarité davantage portée sur le travail. Cependant, certains points retiennent notre vigilance et nous veillerons à ce que les choix qui seront opérés l'année prochaine restent sur la ligne du sérieux budgétaire. La parole

le Président de la République a annoncé son intention de rénover en profondeur le système des minima sociaux afin de permettre une égalité des chances réelles pour nos concitoyens. Cette priorité se traduit cette année par la progression de 6,7 % des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances Cette augmentation est portée par l'évolution de l'AAH, mais surtout par l'accélération de la revalorisation de la prime d'activité. À l'issue de la concertation auprès du grand public relative au revenu universel d'activité, l'analyse parlementaire de cette mission budgétaire revêt un rôle plus que jamais central.

Toutefois, le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit qu'une « augmentation maîtrisée » de 0,3 % de cette allocation. Il convient donc de rester vigilant sur ce point. En effet, il ne faudrait pas que cette sous-revalorisation devienne la norme et déclenche un décrochage du pouvoir d'achat de ces allocataires pour les années à venir. Par nature, l'AAH emporte de nombreuses spécificités. Ainsi, nous sommes très réservés à l'égard de son absorption dans le futur revenu universel d'activité. Concernant le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », il permet de mettre en oeuvre la politique de lutte contre la pauvreté. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d'affecter 9,5 milliards d'euros à la prime d'activité, soit une hausse de 10 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2019 et de 70 % par rapport à 2018. Comme l'a souligné fort justement notre rapporteur pour avis, la prime d'activité est ainsi devenue une dépense majeure de soutien du pouvoir d'achat des travailleurs les plus modestes. De plus, l'augmentation de 52 % de son taux de recours est une très bonne nouvelle. Si nous souscrivons aux objectifs de simplification, le passage au revenu universel d'activité est censé se faire à enveloppe constante. Dès lors, cette hypothèse peut-elle être crédible, si elle s'accompagne d'une augmentation du taux de recours ? Par ailleurs, cette ligne budgétaire traduit également votre ambition pour la mise en oeuvre du plan de lutte contre la pauvreté. Cette stratégie inclut la création d'un service public pour l'insertion et vous lancez actuellement une expérimentation territoriale. Je salue cette initiative qui permet de tester en grandeur nature- et de corriger -un futur déploiement national. Cependant, les départements qui s'y engageront demandent à être rassurés sur un point : ces nouvelles dépenses doivent sortir des « accords de Cahors » qui limitent l'évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an-

S'agissant de la situation des mineurs non accompagnés, je réitère aujourd'hui ma demande d'une vraie prise en charge de cette compétence par l'État en raison des difficultés des départements à y répondre. En dépit de l'augmentation des crédits consacrés à l'accueil des mineurs, le problème réside plutôt dans le fait que les départements n'arrivent pas, d'une part, à proposer des solutions d'hébergement satisfaisantes pour ces jeunes et, d'autre part, à accompagner les psychotraumatismes subis par ces jeunes. Sur ce dernier point, il me semble urgent de multiplier les centres ressources permettant des prises en charge thérapeutiques, individuelles et collectives, ayant notamment recours à des compétences de psychocliniciens. En réalité, les crédits proposés ne sont qu'une aide ponctuelle et ne répondent pas aux problèmes de fond. Enfin, je regrette que le programme 137 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes soit reconduit en 2020 avec un montant similaire à celui de 2019.

près de 15 % de la population française vit en dessous du seuil de pauvreté et ce chiffre est en augmentation. Un enfant sur cinq est victime La France, pourtant sixième puissance économique mondiale, est un pays, où les inégalités se creusent et où les pires injustices côtoient les fortunes les plus insolentes. J'ai souhaité commencer ainsi mon propos, parce que le budget dont nous débattons aujourd'hui doit nécessairement s'apprécier au regard de ces chiffres qui sont autant de parcours de vie faits d'angoisses, de difficultés, de privations, de projets et d'ambitions refoulés, de peur de l'avenir C'est au regard de l'ampleur des urgences sociales et du chantier immense de l'égalité que nous pouvons faire la différence entre ce qui relève de l'aumône ou de la justice sociale, de la charité ou du respect de la dignité. Manifestement, votre budget, au-delà des apparences, n'est pas à la hauteur de la situation et de ces exigences. Je prendrai trois exemples. Vous vous félicitez d'abord de la revalorisation de la prime d'activité, alors que celle-ci n'est qu'un cache-misère social. Les « gilets jaunes », auxquels vous avez notamment répondu par cette prime, et plus globalement toutes les travailleuses et tous les travailleurs de ce pays

faire, vous maintenez le SMIC à un niveau trop bas et vous soutenez les entreprises dans leur politique de régression salariale, en leur accordant des exonérations et allégements de cotisations sociales sur les bas salaires. La prime d'activité, même revalorisée, est insuffisante pour augmenter significativement le pouvoir d'achat. Contrairement aux augmentations de salaire, elle ne concerne pas tout le monde, mais surtout, elle est financée par les salariés eux-mêmes C'est bien à ce tour de passe-passe que nous assistons, quand vous ne compensez pas le coût des exonérations de cotisations sociales pour la sécurité sociale. Deuxième exemple : la revalorisation de l'AAH. Je souligne Je souligne tout d'abord que la revalorisation à 900 euros par mois, montant qui reste en dessous du seuil de pauvreté, n'est pas une mesure exceptionnelle et qu'elle aurait dû être prise il y a déjà plusieurs années pour compenser l'augmentation du coût de la vie. vie. Surtout, elle est en partie annulée par le durcissement des règles de calcul pour les personnes vivant en couple : 67 000 allocataires sont concernés. Nous tenons à réaffirmer notre opposition à la prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l'AAH, comme nous l'avions signifié dans notre proposition de loi qui, malheureusement, n'a pas été adoptée. pas été adoptée. L'AAH est un droit individuel censé garantir l'autonomie de la personne en situation de handicap, quelle que soit sa situation familiale. La règle actuelle est non seulement pénalisante financièrement, mais très discutable sur le plan moral et humain. Elle est aussi parfois vécue de façon infamante par des personnes placées ainsi en situation de dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint. Sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est mon troisième point, la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » n'est pas au niveau. La grande cause du quinquennat qu'est l'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes, ne se traduit toujours pas budgétairement. Pis, les crédits pour le programme 137 sont en baisse, contrairement à ce que vous laissez entendre dans vos déclarations publiques. Votre gouvernement est loin d'être à la hauteur de la mobilisation exceptionnelle de nos concitoyennes et de nos concitoyens sur la question des violences faites aux femmes. Les associations sont extrêmement déçues à l'issue du Grenelle : beaucoup de bonnes intentions, certes, mais quels moyens humains et financiers pour les mettre en oeuvre ?

Des résultats qui, ici, ne sont ni plus ni moins que des vies humaines à sauver, des femmes en danger auxquelles il faut porter assistance et qu'il faut protéger. Il est bon de se le rappeler en permanence. Nos concitoyennes et nos concitoyens attendent beaucoup plus que des demi-mesures. Ils sauront le rappeler utilement dès le 5 décembre à l'occasion des grèves et manifestations contre la réforme des retraites. Pour toutes ces raisons, le groupe CRCE ne votera pas les crédits de cette mission.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, s'il y a un domaine, où l'effort de la Nation ne doit pas faiblir, c'est bien celui de la solidarité. Les crédits de cette mission augmentent de 6,7

qui permet d'accompagner le nombre croissant de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et surtout de la prime d'activité- ces deux dispositifs ont été revalorisés l'année dernière conformément aux engagements présidentiels.

Leur analyse rejoint d'ailleurs les conclusions du portrait social de la France publié par l'Insee le 19 novembre dernier, selon lequel les augmentations de prestations sociales ont fait des gagnants, mais aussi des perdants. C'est toute l'ambiguïté de ce budget, où des mesures populaires voisinent avec des restrictions plus discrètes. Tout d'abord, concernant l'AAH, je souscris je souscris bien évidemment à l'effort budgétaire consenti pour augmenter cette aide sur les deux années 2018 et 2019. Je rappellerai d'ailleurs que notre majorité avait fortement revalorisé l'AAH avait été de 25 %. Cependant, comme je le disais, plusieurs mesures viennent neutraliser la portée de ces revalorisations.

Un quart des allocataires de l'AAH vit en couple ; 40 % d'entre eux y perdront, soit environ 100 000 personnes. À l'image du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, Philippe Mouiller, je déplore la brutalité de cet alignement par le bas de l'AAH. Deuxième coup de rabot, le complément de ressource en cas d'incapacité supérieure à 80 % disparaît pour les nouveaux allocataires. Les calculs montrent une perte pouvant s'élever à près de 180 euros pour les publics les plus précaires, soit entre 7 000 et 10 000 personnes. Enfin, l'AAH n'est pas indexée sur l'inflation pour la seconde année consécutive. En 2020, elle ne sera revalorisée que de 0,3 %. Souhaitons que cette pratique de désindexation qui permet à l'État de faire des économies ne devienne pas systématique ! Je rappelle que, si l'AAH est de 900 euros depuis le 1 novembre 2019, le seuil de pauvreté est de 1 026 euros par mois. L'AAH se situe donc toujours sous ce seuil. Au-delà de ce constat se pose la question de la place de l'AAH dans le futur dispositif du revenu universel d'activité. L'AAH a été créée spécifiquement par la loi de 2005 pour compenser le handicap et l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, souvent de façon irréversible. Ce n'est donc pas un minimum social comme un autre. Certes, le dispositif pourrait gagner en simplification, mais l'absence de visibilité de la réforme inquiète à juste titre les associations. Il vous appartiendra donc, madame la secrétaire d'État, de rassurer les personnes handicapées et leurs familles, comme vous avez pu le faire en partie en audition, en garantissant le maintien des moyens actuels et l'absence de condition d'activité. De même que pour l'AAH, je relèverai quelques déséquilibres dans la répartition de la prime d'activité. Remplaçant l'ancienne prime pour l'emploi et le RSA activité, elle bénéficie largement de l'augmentation des crédits de la mission en en raison d'une montée en charge rapide. La revalorisation exceptionnelle de 90 euros est progressive, et non forfaitaire : les ménages travaillant le moins ou ayant les salaires les plus faibles n'en bénéficient pas. La part de foyers bénéficiaires, dont les revenus sont inférieurs à 1 000 euros, diminue également, elle passe de 41 % à 30 %. Globalement, le public éligible a été élargi au niveau des rémunérations les plus élevées parmi les bénéficiaires et majoritairement à des personnes seules. Enfin, la prime d'activité connaît la même sous-revalorisation que l'AAH- 0,3 % -et n'est plus indexée sur l'inflation. Si un effort est réellement fait en direction de l'AAH et de la prime d'activité, je pense que ces ajustements sont regrettables. Ils créent chez les publics concernés un sentiment d'injustice et d'engagements non tenus. Concernant les autres programmes de la mission, je souhaiterais évoquer les crédits consacrés à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils sont simplement reconduits à l'identique cette année, alors qu'il faudrait mobiliser des financements pour suivre les orientations de cette grande cause nationale du quinquennat. Cette semaine s'est achevé le Grenelle contre les violences conjugales. Cependant, les mesures envisagées- formation, création de postes d'intervenants sociaux, etc. -ne sont pas financées dans le présent projet de loi de finances. Par conséquent, pourriez-vous nous préciser, madame la secrétaire d'État, les modalités de financement qui Au sein du même programme, nos rapporteurs ont souligné que les crédits prévus pour l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle qui est versée dans le cadre de la sortie de la prostitution diminuent pour la deuxième année consécutive. Cette baisse importante- elle est de 40 % -est contradictoire avec l'ambition de départ de la loi du 13 avril 2016 et succède à une série de retards dans la mise en oeuvre du dispositif. Je soutiendrai donc l'amendement proposé par le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, Philippe Mouiller, dont je salue la qualité du travail. J'espère, madame la secrétaire d'État, que vous y serez favorable. Pour conclure, hormis ces réserves, le groupe Les Républicains constate l'évolution positive des crédits de la mission et sera donc favorable à leur adoption dans un souci de protection des populations les plus fragiles. Mes chers